après un engagement de la procédure accélérée d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 77 rectifier au sein de l'article 3.

L'alinéa 7 tend à réduire les obligations de l'employeur en matière de reclassements pour inaptitude et à diminuer les protections légales donc bénéficier les salariés, y compris en ce qui concerne la contestation de l'avis d'inaptitude. C'est bien pour cela que je propose de supprimer l'alinéa cette merci. Merci mon cher collègue, l'amendement identique 121 monsieur Vatrin. Vous le présenter. Une nouvelle fois le gouvernement cède au fantasme que faciliter les licenciements, créer de l'emploi, en effet, en allégeant les obligations de reclassements par l'employeur des salariés rendu inaptes à leur poste, c'est une véritable trappe à chômage qui est créé peut d'ailleurs s'interroger sur les objectifs poursuivis par celui-ci, mais je me doute bien le fait que le 1er motif d'annulation des plantes sociaux par la justice, soit l'absence de plan de reclassements joue un rôle important, car en effet, si le gouvernement cherche à revenir sur cette obligation de reclassements dans le cas des plans sociaux, il ne pourra le faire que dans le cas d'une remise à plat totale des obligations de reclassement, y compris Les mesures dignes la mesure proposée nous semble pas correctes, tant le nombre d'accidents et de maladies du travail régulièrement incapacitants est important malgré un taux de non-déclaration élevé, concrètement, la mesure ne pourra commettre un peu plus une omerta sur les accidents du travail et les Andes incapacité faisant prendre des risques aux salariés concernés, mais aussi à l'école, leurs collègues était le sens de cet amendement de suppression de la ligne. Merci mon cher collègue, l'amendement 42 rectifier Madame Gillot, vous le présenter. C'est sûr que je présente le président monsieur le ministre, chers collègues, la reconnaissance de qualités travailleur handicapé la déclaration d'inaptitude professionnelle sont actuellement une double peine pour le salarié, il subit les conséquences de son inaptitude dans sa vie quotidienne en dehors du travail et dans la très grande majorité des cas, l'avis d'inaptitude est suivi à plus ou moins brève échéance par un licenciement dans son rapport de novembre 2014 sur les Liens entre handicapé pauvreté c'est particulièrement François Chérèque dont je tiens ici à saluer la mémoire et l'engagement, dresse un constat plus qu'alarmant concernant les conséquences de l'inaptitude professionnelle, ce rapport fait écho aux résultats d'enquêtes régionales a donné à des données nationales sur le sujet

dans les avis d'inaptitude rendu comme on peut s'y attendre, les études pointent également une sur-représentation des salariés peu ou pas qualifiés pourcent sont titulaires d'un diplôme infra-Bach ainsi que parmi les plus âgés, 2 populations qui parviennent plus difficilement à reconstruire un parcours de formation dans un autre secteur d'activité, alors il est impératif que nous sortions de ce paradigme de l'inaptitude où les personnes sont jugées, stigmatisées pour ce qu'elles ne sont plus en mesure de faire alors que nous devrions valoriser ce qu'elles sont aptes à réaliser avec leurs capacités restantes développé à développer ou acquérir cet amendement propose une nouvelle rédaction de La Linea cette vague qui propose une nouvelle reine reurs et d'action de la 7 va dans cette direction en permettant à chaque branche professionnelle de définir en son sein les aptitudes recherchées suffisante pour occuper un poste est ainsi valorisé les aptitudes des travailleurs handicapés, leur permettant de conserver ou de retrouver par conversion un emploi dans leur secteur d'activité, cette disposition pourrait également permettre de clarifier les obligations de reclassements de l'employeur et de contribuer à la sécurisation du parcours des salariés. La situation actuelle est inacceptable, il est urgent d'agir pour améliorer le système d'aptitude l'inaptitude professionnelle, actuellement responsable d'un immense gâchis humain votants cet amendement et je suis convaincu que le gouvernement il est partenaires sociaux prendront leurs responsabilités pour que les dispositions en résultant soit utile à l'. Car collègues l'amendement de sens de rectifier terme Madame mourir il vous vouliez la parole. Si Monsieur Président les procédures en matière d'inaptitude à l'emploi sont lourdes et compliquées, il convient de les simplifier. Merci l'amendement 223 présenté par le gouvernement Monsieur ministre ou par le ministre. Oui, pardonnez-moi ce président en 1er lieu déjà pour excuser, madame la ministre, Muriel Pénicaud, qui êtes retenu toute la matinée pour un certain nombre de concertation qui se poursuit avec le 1er Nice et les partenaires sociaux, vous savez nous on nous avons souhaité placer cette réforme hé bien sous sous ses auspices de dialogue et concertation ce qui m'amène aujourd'hui à la suppléé par cet amendement, en fait, le gouvernement souhaite élargir un petit peu les documents prises en compte, donc on ne parle pas seulement des avis, mais également des propositions conclusions écrites ou indication émis par le médecin du travail, voilà, donc je pense que c'est positif et important. Merci monsieur le ministre, quel est l'avis de la Commission, monsieur le président, rapporteur.

défavorable, le 121 c'est le même, c'est donc un avis défavorable de la commission le 42 rectifier c'est un amendement qui pose 3 difficultés sur la forme, il pourrait être perçu comme un élargissement du Champ de l'habitation, ce qui serait contraire à l'article 38 de la Constitution sur le fond, je ne suis pas certain que le niveau d'avant, souhaite adapter pour définir une liste de postes de reclassement pour les salariés inapte, c'est plutôt le niveau d'entreprises qui nous semble pertinent, enfin la nouvelle rédaction proposée par cette amendement écrase notre 10 distinction d'inaptitude d'origine professionnelle non professionnels que nous avions introduite en commission et pour toutes ces raisons, la commission demande un retrait sinon est-ce qu'on voulait mettre un avis défavorable pour l'amendement 211 rectifier terre comme j'avais indiqué à son auteur, la semaine dernière, je ne vois pas ce que la notion de simplification ajoute de plus à celle de clarification, donc la commission ne souhaite pas alourdir le texte nous pensons qu'il reviendra aux parlementaires de vérifier si le gouvernement a rempli ses objectifs de simplification lors de l'examen de ratification des ordonnances, c'est donc une demande de retrait sinon un avis défavorable, mais pour l'amendement 223 du gouvernement, celui-ci souhaite sécuriser les modalités de contestation des avis proposition conclusions écrites ou indication émises par le médecin du travail n'est plus seulement la contestation des avis d'inaptitude, la réforme de la médecine de travail prévu dans la loi travail a en effet précisé la portée de ces différentes notions notamment aux articles L.. 122 6 2 et suivants du Code du travail qui traite de l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnels, donc, la commission est favorable à cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur, je vais donc mettre ou voir. Le Parlement. Merci Monsieur le président, mais le gouvernement a les mêmes avis de la commission donc je vais vous dire exactement ce qu'il en est pour l'amendement 77 rectifier donc un avis effectivement défavorable parce que, en fait, nous souhaitons à me scientiste par cette habitation vraiment examiné toutes les pistes possibles pour permettre au juge prud'homal de prendre sa décision dans des délais plus réduits et des conditions plus optimale et c'est vrai que on on a remarqué qu'un certain nombre de conseils prud'homaux avaient du mal à se prononcer sur les avis médicaux, donc il y a, il y a là un enjeu qui est important pour les salariés comme pour les employeurs, et c'est pour cela que nous ne pouvons souscrire à la suppression pure et simple de l'alinéa que vous proposez, c'est la même argumentation pour effectivement l'amendement 121 de Dominique Vatrin s'agissant de l'amendement 42 rectifier de Madame Gillot. Effectivement, je comprends le souci qui est le vôtre, madame la sénatrice, néanmoins, il nous semble que demander à l'accord de branche, hein, de définir une liste des aptitudes nécessaires peut-être hé bien empêcherait d'avoir vraiment une appréciation personnalisé, sur mesure, or on le sait, dans ce type de situation, il faut tient compte des situations particulières et on aimerait qu'on finalement cette liste d'aptitude, se transformant en compétences minimales en critères minimaux et donc notre crainte est que le mieux sur l'ennemi du bien et donc on comprend la philosophie on y on y souscrit, mais nous pensons à ce stade qu'il convient d'en d'en rester à la rédaction proposée par le gouvernement et la Commission dans le texte que nous discutons et donc c'est une c'est un avis défavorable, s'agissant de l'amendement 211 rectifier terrain présenté par Madame Moret Richot effectivement, je crois, la notion de de simplification elle et dans celle de clarification, finalement, Partage cette philosophie de mettre effectivement de la simplicité, mais la notion de clarification, je crois, permet de prendre en compte pleinement cela et et donc c'est un avis défavorable également

la précision des amendements, c'est de garder des protections légales qui risque d'être mise en cause avec les ordonnances, c'est, c'est une question fondamentale : ça a été abordées aussi bien par Dominique Gillot que monsieur qu'il y a peu de reclassements et qu'on préfère régler les problèmes par un départ de l'entreprise, ces personnes auront connaissent de graves difficultés pour retrouver un emploi et on est dans les trappes à pauvreté. Dans les trappes à pauvreté et c'est pour cela que vouloir garder les protections légales comme c'était demandé dans les amendements est vraiment une bonne solution, je donne un exemple : vous avez vu que la presse économique, titre aujourd'hui sur le résultat exceptionnel de PSA, plus 10,7 pourcent en Bourse. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on passe à des gains de 3 18 pourcent à à 18 66 monsieur Tavarès nous dit fort justement, il faut se féliciter, hein, qu'il y a des des choses comme celles-là qui va couvrir les investissements uniquement par la trésorerie, mais il faut savoir aussi que tout cela a été obtenu par des sacrifices extraordinaires du personnel. Il doit y avoir des embauches et il doit y avoir aussi ce qu'on appelle le salaire indirect, il doit y avoir aussi lorsque, il y a des maladies du travail lorsqu'il y a des incapacités il faut absolument que l'entreprise remplisse ses obligations et si vous diminuez ces obligations, hé bien, toujours, ça se traduira par des licenciements, ça se traduira par pour des personnes qui ne pourront pas retrouver un travail et tomberont dans des trappes à pauvreté, c'est pour ça que faisons attention à ce que nous faisons et je pense que ces ordonnances sont très malvenue, mais surtout, elles vont se tenir sur des questions essentielles dans les villes où nous sommes élus, on va voir la pauvreté augmenter on voir des personnes qui, comment, ont eu des maladies du travail et vont tomber et vont se retrouver au RSA, quelques années après, voilà, c'est pour ça que je soutiens, je pense qu'il faut soutenir

Ces contrôles. Qui s'abstient, ils ne sont pas adoptées, l'amendement 42 rectifier, vous avez la parole Madame Gillot. crois, je reviens sur mon argumentation, alors je comprends qu'. ça peut être. Un peu, un peu difficiles et que la liste des aptitudes demandées à la branche puisse se réduire ensuite. Une liste de compétences minimales qui pourrait être opposé à des à des reclassements, néanmoins, je pense que c'est important de regarder la personne handicapée en fonction de ses capacités en fonction de 6 aptitudes plutôt qu'en fonction de ses inaptitude et l'amendement du gouvernement simplement confié cette responsabilité aux médecins du travail, me paraît être un peu un peu imprudent, surtout compte tenu de la situation de la médecine du travail aujourd'hui, dont on a quand même abondamment discuté et compte tenu de l'inexpérience des médecins du travail sur les aptitudes nécessaires à un reclassements, donc souvent l'avis médical se conclut par une inaptitude au travail qui se conclut par une une un rejet de, de, de, des capacités restantes ou à développer ou que le la personne peut acquérir donc ce qui est important, c'est qu'on ait cette préoccupation est que dans le dialogue social, la parole soit donnée donnée à la personne elle même aux travailleurs, aux salariés pour qu'ils puissent dire quand il est jugé inapte à un point, un poste, et bien qu'il peut être apte à un autre poste dans la même branche dans la même entreprise en fonction des aptitudes restantes et en fonction des aptitudes qu'il peut développer par une formation bien adapté, ou par une adaptation de son poste de travail qui n'est pas forcément coûteuses ou insupportable pour le chef d'entreprise, c'est vraiment un changement de paradigme auquel le je, je, je, que j'appelle parce que sinon, on a 500000 chômeurs on en fabrique 150000 tous les ans et il y a pas moyen de faire rentrer les travailleurs avec handicap dans l'emploi parce que ils sont frappés d'une interdiction de travail à cause de l'inaptitude du classement inaptitude au travail ou reconnaissance de travailleur handicapé qui ne trouve pas sa place aujourd'hui dans le reclassements, donc il y a vraiment un changement de modèle, un changement de paradigme à prendre et il me semble que le dialogue social est le mieux à même pour prendre en considération, alors peut-être que le niveau de la branche n'est pas n'est pas satisfaisant le niveau de l'entreprise doit l'être, mais il faudrait qu'il y a un guide et que on ne s'en remettent pas uniquement à l'avis du médecin du travail qui souvent n'est pas qualifié pour pour proposer des reclassements. Image chers collègue de Madame pour explication de vote. Oui, moi je reconnais beaucoup de cohérence à notre collègue Dominique Gillot dans le la volonté qu'elle a et qu'on a du reste préempte compte il y a ce soir ou cette nuit, au travers de ces amendements, de faire en sorte que, il y a une effectivité à l'égalité des travailleurs handicapés qui soient pris en compte comme des personnes au travail n'est pas d'abord comme des handicapés, mais je pense que, compte tenu aussi de ce que nous avons voté, à l'article 1 qui est quand même fondamental pour le coup c'est l'articulation entre la branche et l'entreprise et donc on a élargi, de ce fait, le Champ de la branche et je crois que là c'est typiquement puisqu'il s'agit de, de, de postes de travail, c'est typiquement du ressort du niveau de l'entreprise parce que il faut prendre en compte le secteur d'activité, ça me paraît le plus le critère le plus essentiel et actuellement les branches, là aussi, on a voté un homme, un amendement du gouvernement avec l'accord de la Commission, qui réduit le délai dans lequel les branches doivent se restructure et je rappelle qu'elles sont 650 aujourd'hui que nombre d'entre elles ne correspondent plus à des métiers et encore moins des métiers de demain, donc je pense qu'il faut prendre en compte cela et c'est vrai que le dernier argument que je voudrais vous convaincre Madame Gillot, c'est par rapport à la médecine du travail, on sait que c'est une médecine en carence madame la ministre, hier soir, a dit qu'effectivement il fallait demander du reste un rapport à l'IGAS, qu'elle doit avoir, à la fin du mois de septembre, je crois, et il faudrait effectivement que la médecine du travail à partir de là soit réformé et que on lève le le vrai problème, c'est-à-dire l'absence de et il attractivité de ce métier de médecin du travail donc ça fait partie de des préoccupations du gouvernement et ça fait partie des nôtres, rappelez-vous les débats pose allongée sur la loi dite El-Khomri donc voilà, moi, j'essaie de convaincre et de comprendre l'argumentation, plutôt que de ne pas l'écouter comme ça arrive sur certains amendements. Par collègues Madame Génisson pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, c'est un moment et et et très intéressant et et nous allons le le voter, je crois qu'au-delà des explications qui viennent d'être donnés, et en particulier celles qui comment dire dans la course, le médecin du travail, il faut se dire qu'au-delà de tout, tout ce que l'on peut faire en matière d'appréciation d'aptitude, il y a toujours l'adéquation entre le poste proposé et l'appétence du salarié a occupé de ce pour ce poste, et ça c'est vraiment le colloque singulier entre le médecin du travail et et le salarié concerné, je crois qu'il faut jamais perdre ça de il faut toujours garder ça à l'esprit et ça me semble très, très important et ça permet bien évidemment de insister sur le sujet de la médecine du travail et la carence en la matière dont nous sommes tous collectivement coupables. Merci, ma chère collègue Monsieur Savary pose plus question de vote. il faut bien différencier les causes et les conséquences de l'inaptitude parce qu'il y a des causes qui peuvent être des causes liées au travail, avec des conséquences sur l'inaptitude bien sûr au travail mais des causes liées à la vie domestique, un accident sportifs etc qui font que, derrière, il y a une petite inné inaptitude au travail. Donc c'est pas, me semble-t-il systématiquement à l'entreprise de prendre en compte toute la gravité de l'accident ou de la maladie, selon l'imputation qu'on peut lui faire sur le plan de l'origine de la pathologie, d'autre part, les reclassements sont différents, si on appartient, une petite ou une grande entreprise dans une grande entreprise il y a quand même un éventail relativement large dans une petite entreprise, le reclassement et un peu plus contraint la réflexion autre branches. Et entreprises, a également ses limites parce que quand on est qualifié dans une branche, il n'y a pas forcément des entreprises de cette branche, qui sont dans le même bassin d'emploi, donc l'ordonnance doit permettre d'avoir une réflexion par bassin d'emploi, ce qui serait important pour prendre en compte véritablement cette personne dans le cadre de son intégration locale, ce qui est très est intéressant, c'est de voir comment l'échelle ou de Pôle emploi ou d'autres, on puisse travailler un reclassements dans le bassin d'emploi, avec des actions de formation pour prendre en compte cette personne dans son lieu de vie et maintenant la télé-médecine du travail, une avancée quand même qui a été signifié de par la loi, même si on a, on verra les résultats l'évaluation que dans quelques années la télé-médecine du travail permet localement au niveau des bassins d'avoir une vision des types d'emplois qui assure un bassin d'emploi et de mieux reclasser les personnes en difficulté donc j'invite le gouvernement dans le cas de ces ordonnances a véritablement travaillé toutes ces pistes et on aura un progrès qui sera fait à ce moment-là, sur la prise en compte des gens qui connaissent ces problèmes d'inaptitude. sur ce sujet du handicap et de la prise en compte effectivement de de ces situations très clairement, je je veux rassurer sur le fait que nous prenons en compte le gouvernement souhaite prendre en compte cette dimension le 3ème plan santé au travail, vous le savez, a été discutée il y a peu, il comprend un volet justement qui qui qui qui aborde naturellement au fond et et qu'il y a, il apporte des réponses également justement pour lutter contre la désinsertion professionnelle et notamment sur ce volet des des personnes handicapées, c'est un plan qui d'ailleurs a recueilli l'assentiment de l'ensemble des partenaires sociaux, encore une fois, apportant des réponses et et donc ça soyez vraiment assurer notre détermination à dans la vie concrète et réelle, être aux côtés de ces personnes, effectivement, et notamment dans ces situations, mais c'est vrai que, en terme d'écriture de de de cette loi et,

je vous demande votre compréhension sur le fait que nous soyons défavorable à cet amendement et je remercie par ailleurs Madame Bricq, pour ces précisions et René-Paul Savary pour les perspectives quittera sur des sujets qui sont effectivement un petit peu distincts mais qui sont vraiment très importants par rapport aux notions de territoire.

je voulais à ce stade, indiqué que dans les petites entreprises en cas d'inaptitude, on a souvent malheureusement pas de poste à proposer et cette inaptitude peut entraîner un licenciement Monsieur le ministre, dans certains cas, donc les employées ont une ancienneté le licenciement peut, ça peut s'avérer extrêmement lourd et en coûte bien sûr, même si bien sûr c'est très embêtant pour la personne qui va être licencié, mais peut s'avérer très lourd en coûte pour l'entreprise et l'entreprise peut-être obligés prenait pour licencier, ça m'est arrivé dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, je pense que si vous voulez l'inaptitude et ça ne devrait pas être entraîné de coûte à l'entreprise, c'est pas de la faute de l'entreprise, si la personne est inapte et c'est pourtant l'entreprise qui est pénalisé, donc je voulais Monsieur le ministre vous indiquer cela merci. Merci mon cher collègue, monsieur Laménie pour explication de vote. Oui merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, concernant ces amendements, je comprends tout à fait ces questions un sujet particulièrement sensible de la médecine du travail de l'inaptitude mais aussi du du handicap parce que il faut le reconnaître aussi dans nos départements respectifs, nous avons aussi les ESAT, ce qu'on appelait aussi les ateliers protégés, donc il y a aussi des personnes qui travaillent aussi pour le monde économique, industriel, notamment en sous-traitance et je crois que c'est aussi parallèlement, on sait aussi qu'il y a un manque de, de postes de place aussi à ce niveau-là, bon c'est c'est d'autres Budgets mais je crois que tout est étroitement lié, parce que je crois que l'activité économique, c'est toutes les personnes je dirais toutes les catégories à prendre en compte avec de, de, de, d'accessibilité discernement aussi il faut le dire et et beaucoup de respect, je crois que, à tous les niveaux, je crois que chacun utile et je crois, il faut essayer aussi de de répondre aux attentes et je crois que c'est aussi un volet utile fortement il y a, on sait aussi que passés amendement c'est peut être aussi une certaine manière, des amendements d'appel pour faire évoluer les choses positivement voilà dans le sens du dur de la commission des affaires sociales, Jean merci. Merci mon cher collègue, je vais dans mettre ou voile amendements 42 rectifier il y a 2 avis défavorables qui est pour cet amendement. Qui est contre. Qui s'abstient l'amendement n'est pas adopté, nous arrivons à l'amendement 200 rectifier et vous aviez une demande de retrait Madame Maury riche. Merci monsieur le président. J'ai bien entendu donc le la vie de notre rapporteur et aussi je retire l'amendement. Oui, ma chère collègue et nous arrivons à l'amendement 223 du gouvernement avec un avis favorable de la commission qui est pour, pardon, Madame Gillot, vous avez la parole.

simplement, je voudrais vous quand même que vous soyez tous conscient dans cette salle, dans cet hémicycle, qu'une personne handicapée veut être considérée par rapport à ses aptitudes, pas par rapport à son handicap, quelles que soient les conditions d'acquisition de ce handicap, que ce soit dans le milieu du travail dans le milieu domestique dans le milieu sportif, la personne qui devient handicapée qui vit avec son handicap, elle le dépasse, elle puise au fond d'elle-même des ressources les aptitudes des facultés qu'elle aurait laissé en jachère, si ça n'avait pas été le cas équipe est une chance, une possibilité de reconstruire sa vie, or aujourd'hui on considère le travailleur handicapé comme une obligation de reclassements comme un poids pour l'entreprise et pour la société, essayons de de changer de regard, de changer de paradigme et disons-nous qu'une personne qui a, qui a un handicap, hé bien elle a acquis des compétences, elle est capable de dépasser tout ça d'organiser sa vie c'est un Manager c'est une voilà c'est des personnes qui ont une force de vie, une force de travail qui est très intéressante, à la fois pour l'entreprise et pour la société, donc je pense qu'il est très important qu'on change le regard qu'on change le, la manière de considérer la personne handicapée, même au travail, ce n'est pas un boulet, ce n'est pas une contrainte, c'est une personne qui a des compétences, qui a des aptitudes à mettre au service de la collectivité et des autres. Merci la charte, je vais donc. Bonjour à l'amendement 223 du gouvernement avec un avis favorable de la commission qui est pour cet amendement. Est contre cet amendement, l'amendement est adopté, nous arrivons à 3 amendements qui font l'objet d'une discussion commune, devançant même de monsieur Vatrin, vous avez la parole. Oui, la lignée numéro 10 de cette article prévoit de faciliter le recours au départ volontaire dans le cas des plans de licenciements, nous demandons que cette facilitation soit abandonnée en effet si les plantes départs volontaires peuvent être conçue comme une alternative aux licenciements secs leurs DPS ce cette alternative n'a pas les mêmes conséquences pour les salariés, ainsi, alors que les licenciements obéissent au cadrage légal du PSU Les départs volontaires sont le fruit de négociations avec l'employeur, qui peuvent être donc moins favorable, bien sûr, ces plans peuvent dans certains cas, répondent aux aspirations de certains salariés, personne ne le niera, mais ces dispositifs existent déjà et rien ne justifie de les faciliter plus encore, comme il est proposé ici inscrire dans le code du travail, la simplification de cette démarche, cela revient à casser les protections aujourd'hui offerte aux salariés, monsieur le ministre avait répondu à nos collègues de l'assemblée qui vous présenter les mêmes réserves à cette pratique et vous avez répondu qu'elle résulte d'une combinaison d'articles du code du travail du Code civil et la jurisprudence du coup les obligations qui en découlent ne sont pas l'toujours lisibles et par conséquent pas sécurisé, ni pour les employeurs, ni pour les salariés, la clarté du droit permet un meilleur exercice du droit pour les 2 parties s'étaient donc la réponse de Madame la ministre devant l'Assemblée nationale, mais en l'espèce, cette clarification bénéficiera bénéficiera surtout aux employeurs de même façon que la logique d'ensemble de ce texte en facilitant le recours aux plantes, départs volontaires vous n'apportez aucune garantie supplémentaire aux salariés tandis que vous permettez aux grandes entreprises de tailler dans leur masse salariale à moindre frais, de quel côté était le volontariat, la liberté de choix quand la direction d'Orange, France Telecom a annoncé ses plans de départs volontaires après avoir instauré un climat malsain au sein de son de l'entreprise, le 20 juin dernier Véolia annoncé vouloir séparer de près de 600 salariés dans sa branche eau d'ici à 2020, précisant qu'il s'agirait là encore départs volontaires, mais il est difficile de croire que ces 600 personnes et tout un projet pour se relancer, pourtant ils ne bénéficieront pas des avantages d'un plan de sauvegarde de l'emploi, telle est le sens de cet amendement. Qui c'est qui le présente Madame Richaud. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le but ici dans cet amendement serait de faciliter le recours au plan de départs volontaires, même pour les TPE et PME qui n'ont pas de représentant du personnel. également, oui, les plans de départs volontaires doivent être envisagées dans le cadre d'une procédure simplifiée, dans l'intérêt des parties. Il y avait de la Commission, monsieur le rapporteur. Sur ces 3 amendements. Monsieur le Président, pour ce qui est de l'amendement 122 présenté pendant entre collègues Vatrin la commission émis un avis défavorable, elle pense qu'il est nécessaire de clarifier le régime juridique des plans départs volontaires qu'on lui applique quasiment systématiquement les règles du licenciement économique, même si aucun licenciement n'est prononcé, in fine, et pour l'amendement 173 rectifier terre la Commission pense que dans les petites entreprises, des plans de départs volontaires n'est pas adapté l'employeur et le ou les salariés concernés ont plutôt tendance à conclure une rupture conventionnelle, qui est un dispositif qui ne semble plus souple que le plan départs volontaires, c'est donc une demande de retrait sinon un avis défavorable, et pour le 173 172 pardon rectifier terre, là encore, nous pensons que l'objectif de simplification du plan départs volontaires et largement satisfait pas celui de sécurisation, mais on ne souhaite pas ajouter systématiquement dans le texte, l'objectif de simplification pour ne pas alourdir celui-ci évidemment et parce que la Commission pense que le gouvernement y souscrit, comme nous le souhaitons, donc ce sera une demande de retrait sinon un avis des Merci monsieur le président, le gouvernement et mais également les mêmes habits que que la commission 3 avis défavorables, peut-être pour apporter une réponse commune finalement à Dominique Vatrin et en même temps à à Patricia maréchaux, en fait, vous l'avez souligné les plantes départs volontaires sont beaucoup issus en terme de de modalités d'une construction jurisprudentielle et donc le fait d'ailleurs d'inscrire c'est PDV dans dans le texte de cette loi et puis donc, dans une ordonnance, fait d'ailleurs qu'on va du coup mettre au niveau législatif, un certain nombre de principes de clarification et quelque part une forme de sécurisation qui devrait je pense vous intéresser et et et gravé dans le marbre de la loi, c'est un nombre d'éléments importants. Et en même temps, madame Moret Richaud, le fait de réunir justement un certain nombre d'éléments pour l'instant éparses, dans des arrêts dans différents codes dans une même ordonnance va apporter de la simplification, celles que vous appelez de vos voeux et que nous partageons et donc s'agissant de du dernier amendement que vous avez présenté sur le notamment pour les TPE-PME Le notamment voilà signifie bien que ces prises en compte, elle, si elles le souhaitent, elles peuvent naturellement avoir recours à ce dispositif, même si le président Millon a souligné à juste titre que d'autres dispositifs pouvaient être plus facile facile à mettre en oeuvre pour leur part, donc 3 demandes de retrait à défaut : avis défavorable Monsieur Président. Monsieur le ministre, je vais mettre au voilà Mandement sans 2 avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient l'amendement n'est pas adopté, je vais passer l'amendement 173. Et puis les Terres et vous êtes sollicité pour en retrait Madame Moret Alors effectivement entendu les différents éléments dément du de la du par date d'une part de la Commission et puis d'autre part du gouvernement, je retire cet amendement. Même chose pour le 2ème madame, Lamure vous avez la parole. Merci monsieur le président, moi je pense que il n'est pas anodin de vouloir introduire de la simplification dans les procédures parce que la simplification, tout le monde en parle, mais on peut noter qu'il y a pas beaucoup de mises en Oeuvres, nous avons auditionné il y a 2 jours, le ministre de l'économie, qui nous a indiqué qu'il ferait de la simplification, la clé de voûte de son action pour la modernisation de notre économie, donc je pense que nous sommes vraiment là dans le sujet et il serait intéressant qu'à tous les niveaux on prenne en compte ce cette volonté de simplification. Merci, ma chère collègue Madame Maury Show sur 172 rectifier terre. Sur cet amendement, donc, en espérant que que la simplification soit effectivement effective dans cette attente, je retire l'amendement si. Nous passons à 16 amendements qui font l'objet, pardon, d'une discussion commune. L'amendement. Je vous en prie, mes chers collègues quinze rectifier bis qui est présenté par Madame Lienemann. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, je propose par cet amendement avec bon nombre de mes collègues, socialiste de supprimer les alinéas 11 à 17 les mesures qui sont indiqués dans ces alinéas sur une véritable prime aux délocalisations, pourquoi, parce que, avec ce mécanisme et et c'était déjà pas brillant Kant le texte nous venait de l'Assemblée nationale, force est de constater qu'il a été encore plus rendu comment antisocial et antiéconomique parlez-vous les votes de notre commission

jusqu'à présent, et notamment une jurisprudence avait de la Cour de cassation l'avait confirmé : on prenait en compte non pas le périmètre sur le territoire national de 10 entreprises d'un même groupe, on prenait la situation économique du groupe globalement c'est un vieillard et puisque c'est un art et vidéo que lors de la cour de cass de 1995 et cette philosophie, elle est fondée, elle est fondée dans une mondialisation où on peut pas considérer que les profits sont captés pour être emmené à l'étranger, tandis que les juges chargés sociales et les conséquences sociales sont portés à l'intérieur du simple payer France d'autre part, on connaît bien, qu'il y a des tas de possibilités de contourner à travers ce genre de mécanisme de faire payer au pays le départ d'entreprises vers l'étranger, comment on fait, prix de transfert. On a dit qu'on fait passer par le mécanisme des prix de transfert des profits et de la de la richesse produite dans une entreprise en France, on le fait passer sur un dans un autre territoire Pierre Body. Que c'est dramatique, l'entreprise n'est pas rentable et et puis ensuite, petit à petit, de fil en aiguille, on vide ses entreprises de leur capacité à produire de la richesse et au débat, il faut licencier, pas assez performant, pas assez compétitifs et on licencie et qui équiperont la charge de fait des conséquences sociales de ça c'est la France, j'y vois donc 2 effets, on accélère les possibilités de préparer des délocalisations et on accélère l'optimisation fiscale parce qu'ils ont maintenant tout intérêt à faire ça, vu que on ne on leur remettra pas, c'est une injure à leur profit globaux. Merci, ma chère collègue l'amendement identique 78 rectifier Biesme scientiste, vous avez la parole.

les conditions d'appréciation des difficultés de l'entreprise et en allégeant les obligations de reclassements, un autre cet alinéa rend possible une modification des critères d'ordre des licenciements ainsi que n'aménagement des seuils à partir duquel les ruptures de contrat de travail sont considérés comme des licenciements collectifs, en fait, il permet d'élargir les possibilités de licencier en cas de cession d'entreprise cet alinéa tend à accroître la précarité du travail, c'est pourquoi nous en proposons la suppression, d'ailleurs,

le gouvernement entend assouplir l'ensemble du droit de licenciement économique, aujourd'hui ça été rappelé les difficultés économiques d'une entreprise ont apprécié au niveau du groupe à l'échelle internationale, le projet de loi permettrait que les difficultés économiques entreprises s'apprécie sur le seul territoire français même si le groupe auquel elle appartient est en bonne santé financière au niveau international, on connaît beaucoup de groupes, effectivement, qui sont dans ce cas-là, en outre, donc cet article prévoit de simplifier le médiation de reclassements, modifier les critères d'ordre de licenciements ainsi que les seuils à partir desquels les ruptures de contrat de travail sont considérés comme des licenciements collectifs qui oblige les entreprises donc à négocier un plan de sauvegarde de l'emploi, enfin en facilitant les possibilités de licenciement en cas de cession d'entreprise cet alinéa remet également en cause les protections légales dont bénéficient les salariés licenciés économiques pour la rédaction de la commission des affaires sociales, c'est en fait une transcription de cette volonté, c'est la raison pour laquelle donc nous en demandons la suppression. Oui, mon cher collègue, l'amendement 165 Madame Bouchoux, vous avez la parole. Monsieur le président, monsieur ministre que je salue Monsieur le Président, la commission monsieur rapporteur, mes chers collègues, nous défendons également la suppression des aléas 11 à 17 et je ne vais pas reprend les excellente démonstration de mes 3 précédents collègues moi en rentrant hier soir j'ai essayé de regarder un petit peu au niveau de l'économétrie ce que donner un petit peu les choses dont nous parlons et je repose à nouveau à monsieur le ministre la question : quelles sont les études économétriques international qui nous montre que ce que nous avons hier soir détricoter du point de vue de la micro-entreprise et ce que nous faisons, ce matin, du point de vue de la facilitation des licenciements en modifiant pour faire simple et périmètre comme l'a dit Marie-Noëlle Lienemann, en quoi cela va créer des vrais emplois à temps plein pérenne pour les travailleurs qui sont en France, pardonnez-moi, mais ce que nous sommes en train de faire et je le dis en tant que franco-allemande en tant que professeur d'économie, que j'ai été que je serai à partir du 1er octobre prochain ce que nous sommes en train de faire, c'est ni plus ni moins, mais 20 ans plus tard, et à mon avis moins bien que les employes rare en Allemagne, c'est uniquement ça, c'est-à-dire que nous allons faire des travailleurs pauvres, précaires dans les services en considérant que tout peut être externalisées et c'est ce processus qui est en train d'être mis en place et de ce fait, il ne nous semble absolument pas rassurant de voir ce qui a été prévu et notamment, comme l'a dit Marie-Noëlle Lienemann, de voir que ça va être la double peine, c'est-à-dire que les entreprises a été vue dans les rapports Bocquet un et 2, que nous avons collectivement validé les entreprises font massivement de l'optimisation fiscale évite les impôts ici en 3 clics avec ça a été bien dit par les prix transfert arrive à fictivement rendre leur situation en France moins confortable moins périlleuse et d'un côté il ne paye presque pas d'impôts et en plus, on va pouvoir licencier plus facilement des salariés, pardon, mais ce que nous sommes en train de mettre en place, ce sont des clés qui est qui dans le contexte de la mondialisation telle qu'elle est actuellement, va nous fabriquer pour 30 ans des travailleurs pauvres s'en protéger, ce ce que l'on emploie et sans créer de manière durable des emplois et je comprends bien que les conditions que nous avons décrit hier soir et maintenant peuvent inquiéter certains chefs d'entreprise qui dit je ne peux pas embaucher si je ne sais pas, que je pourrais licencier facilement, mais je demande de nouveau des preuves scientifiques de cela, nous ne les voyons pas, y compris lorsque nous regardons l'économie allemande, merci.

et cher collègue actuellement les difficultés économiques d'une entreprise qui licencie sont appréciés au niveau du groupe à l'échelle internationale, l'article 3 et je ne crains permettrait de les apprécier sur le seul territoire français même si le groupe auquel elle appartient est en bonne santé financière au niveau international, or, Madame la Ministre, l'a reconnu, lors des débats à l'Assemblée nationale, une minorité, je dis bien une minorité d'entreprises pourraient utiliser une disposition de ce type au créer artificiellement des difficultés au niveau d'une entreprise dans le seul but de justifier les licenciements pour motif économique, c'est pourquoi nous vous proposons de supprimer cet alinéa 12. Si mon cher collègue, la demande de sens 18 rectifier milice. Qui est identique présenté par monsieur Assouline. Oui amendements identiques donc avec cet alinéa 12 ans on revient sur un débat qu'on avait au moment de la loi El-Khomri et heureusement le curseur était bien tomber à ce moment-là, donc il s'agit de remettre cette question pourtant. C'est une des questions sensibles où tout le monde avait pu apprécier qu'il fallait pas se lancer dans cette aventure, parce que ce serait effectivement comme l'a dit Marie-Noëlle Lienemann, une prime aux délocalisations, la Cour de cassation avait réussi à développer une jurisprudence protectrice éclair

au niveau international, ce qui connaissent comme nous tous un petit peu le monde des entreprises ne sont pas sans savoir que quelques multinationales savent habilement mettre leurs filiales françaises dans le rouge et accumuler leurs profits dans des pays où les taxations sont moindres, on nous invite à être dans les travaux pratiques et dans le concret, ça c'est du concret, c'est ce que l'on peut vérifier ce que l'on peut voir, donc il faut s'en prémunir,

la ministre a expliqué à l'Assemblée qu'il s'agissait de mieux définir le périmètre du licenciement économique en proposant une telle définition mais le risque est que le périmètre qui ressortira de cette de ces ordonnances soient si restrictif qui laisse toute latitude aux entreprises pour manier des montages artificiels tout en privant de marge de manoeuvre, juge à l'inverse, si cette définition madame la Libye ministre être était trop vague, elle pourrait remettre en cause la jurisprudence sans apporter de sécurité juridique supplémentaire donc avec cet alinéa, le groupe, nous comprenons que peut-être on veut envoyer un signe aux investisseurs étrangers, mais on sait qu'ils sont déjà à la hausse, c'est pas là qu'il aurait un gros sujet je conclus en disant que dans cette liberté que vous souhaitez accentuée pour les investisseurs, encore une fois, on voit que l'attention de cette loi n'est pas dirigée vers les salariés. Mais toujours vers les mêmes Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre. Il s'agit effectivement il s'agit de La Linea 12 sur lequel la Commission a apporté des restrictions cantonnant le périmètre à l'État à la nation. La rédaction du rapporteur. Préjuge encore une fois des résultats de la concertation avec les partenaires sociaux, il est surtout évident que la rédaction de notre rapporteur, a pour but de revenir sur une jurisprudence de la Cour de cassation, ceci a été souligné qui exige de prendre en compte la diversité des situations des entreprises pour retenir un même périmètre national européen ou mondial, nous avons tous en mémoire des cas de LBO ou la trésorerie des entreprises a été délibérément asséché pour financer d'autres reprises dans un système de cavalerie mondialisé, nous avons vu aussi des groupes cesser tout investissement dans une filiale française pour investir dans d'autres pays, sur d'autres continents. Pas nécessairement sur des marchés plus porteurs parce que pas encore saturé, mais tout simplement pour ne pas avoir à rémunérer une main-d'oeuvre dépourvus de tous droits économiques et sociaux. Quitte à faire revenir ensuite la production en Europe, où se trouve encore des clients solvables grâce à des coûts de transports réduits mais une empreinte carbone élevé en tant qu'élus locaux, en tant que représentant des territoires de la République, nous avons tous eu à traiter des problèmes économiques et des difficultés sociales qui résultat m'encadrement de ces comportements de prédateur, nous avons moi-même sans qu'il soit besoin de prendre en compte ces manipulations en vue de créer des difficultés une filiale française dans un groupe multinational, la prise en compte de la situation globale du groupe doit demeurer un élément d'appréciation de la réalité des difficultés économiques, au-delà de la seule question économique, c'est un aspect, un aspect de la souveraineté nationale qui est en cause, considérez-vous que notre justice est légitime à prendre en compte les agissements d'un groupe qui national sur notre territoire, à mesurer ses agissements à l'aune des profits réalisés grâce à eux, avons-nous le droit de sanctionner des agissements qui, sans être même délictueux sont délibérément préjudiciable à notre économie et à nos citoyens, la et la réponse à cette question semble aujourd'hui négative de votre point de vue pourtant les conséquences économiques, sociales évidemment politique de cette soumission sont déjà bien présentes, il est plus que temps de s'en inquiéter. Merci beaucoup monsieur le président, en fait, par cet amendement, le gouvernement, même s'il partage le souci effectivement d'avoir cette réflexion sur le périmètre ne souhaite pas que on la tranche définitivement ce matin puisque justement, très clairement, il y a un certain nombre, vous le savez, de concertation, qui sont eux en cours, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis devant vous ce matin puisque le ministre est présentement avec les partenaires sociaux et

et donc la rédaction qui vous est proposé est une rédaction qui propose justement de de dire que l'ordonnance définira le périmètre géographique et le secteur d'activité,

Vous le savez, sur une réforme majeure, on le voit bien des attentes très fortes des différents partenaires sociaux patronaux comme syndicaux et et je crois qu'il faut laisser aussi ce temps du dialogue pour que, hé bien il puisse y avoir des décisions qui soient les plus partagés possible et c'est pourquoi le gouvernement propose de revenir. à la rédaction, qui était la sienne, tout en en comprenant bien les préoccupations qui ont été émises par la commission voilà, telle est l'objet de de cet amendement de son président.

pas jeune, en consacrant cette jurisprudence théoriquement quand on licencie pour motif économique au regard de la situation économique de l'entreprise au moment où on licencie l'arrêt PagesJaunes était intéressant puisqu'au moment du licenciement, la société se portait bien, mais elle a évoqué des difficultés économiques objectivement prévisibles, ce qu'elle pouvait prouver les tribunaux ont accepté la démonstration, il faut insister sur le fait qu'il est possible de licenciés économiques avant qu'il ne soit trop tard et que la situation économique ne soit dégradée de manière irréversible, telle est l'objet de cet amendement.

Monsieur le président, Monsieur le ministre, il s'agit de, de, d'une correction d'une précision rédactionnelle en supprimant le terme comptable, alors que si le l'aspect comptable n'est qu'une constatation de la réalité, qu'elle soit artificielle ou non, donc ça c'est le 63 est le suivant, qui est une 2ème proposition parce que je voulais savoir le le la vie un petit peu du du gouvernement et de et de l'Assemblée sur sur ce sujet-là, la 2ème proposition c'est de être artificiel, notamment en termes de présentation comptable pourquoi notamment, c'est-à-dire je demande une modification mon amendement suivant, parce que si on met artificiel en termes de présentation comptable, on ferme, je dirais le le l'aspect artificiels uniquement à une pratique comptable qui ne serait pas vertueuse, donc en mettant artificielle, notamment en termes de présentation comptable, on insiste sur cet aspect d'une comptabilité, on va dire, mais on ne la ferme pas uniquement à cette possibilité, donc c'est c'est une précision parce que mettre uniquement aspect comptable con mais où ça ne veut pas dire grand chose, la comptabilité une quelconque constaté des choses réelles ou des choses qui ont été éventuellement détournés ou falsifiés, mais ce n'est qu'en constat donc on peut pas mettre que l'origine soit comptables. Madame Cohen. Vous avez la parole Madame David excusez-moi. La fatigue, monsieur le président, mais chers collègues par cet amendement 123, nous proposons de rédiger différemment la alinéa 14 de cet article, puisqu'en effet au aujourd'hui nombre des propositions d'Eureco reclassements sont faites à minima pour répondre à une obligation légale sans brut aboutissements réels envisager donc cet amendement vise à renforcer les obligations de l'employeur concernant la crédibilité et le sérieux des offres de classement, nous avons toutes et tous sont têtus mais chers collègues malheureusement des cas comme polymère à La Barre Thomas comme Karmann à Castres, les Fralib de j'noces ou encore Continental de les offres d'emplois qui ont été faites aux salariés de ces entreprises, notamment les offres de reclassements en Pologne, en Roumanie ou encore en en Tunisie était plus une insulte faite aux salariés que de véritables offre de reclassements, pourtant ces offres sont vitales pour les salariés licenciés, cet amendement vise donc à renforcer les exigence de maintien de nos concitoyennes et concitoyens dans l'emploi tout en prenant en compte les réalités économiques des entreprises visées nous tentons nous souhaitons par cet amendement de qualifier ces propositions de reclassements afin de sécuriser quelque peu les salariés licenciés. Si ma chère collègue de l'amendement 175 rectifier Taher Madame Maury Show. Oui, l'objectif est également de sécuriser l'obligation de reclassement à laquelle sont tenus, les chefs d'entreprise cette mention doit on doit donc être inscrite dans la loi. saisit rectifier terre. Les ce que l'on peut dire, c'est que la procédure de licenciement et compliqué et donc il convient de la simplifier, c'est l'objet de cette amendement. Merci, ma chère collègue le 65 actif est

Oui, merci Monsieur le Président, alors pour ce qui est de de l'amendement 15 rectifier bis, la position de de la commission et cohérente, nous souhaitons que le périmètre national soit retenue pour apprécier la cause économique d'un licenciement, et en même temps pour éviter les détournements par des groupes mal intentionnés, nous acceptons l'habilitation demandée par le gouvernement pour détecter les difficultés économiques artificiel ou comptable, notre position, vise à mettre fin à une exception française en Europe car notre législation pendant des années n'a pas défini la notion difficultés économiques a conféré au juge un rôle important pour pallier ce vide juridique, notre position est un compromis : nous ne retenons pas le critère de l'entreprise ni celui européen ou mondial du groupe notre position, vise à renforcer l'attractivité de notre économie, car les investisseurs ne doivent pas se sentir Monsieur le ministre, prisonniers de leurs investissements en France enquête difficultés, c'est donc un avis défavorable pour cet amendement ainsi qu'aux amendements 15 rectifier bis 78 rectifier bis 124 et 165 qui sont identiques à celui-ci, pour ce qui est de l'amendement 196 la commission d'affaires sociales Monsieur Président à modifier la rédaction de la ligne à visé par cet amendement de suppression afin de préciser que c'est bien le périmètre national qui doit être retenu pour apprécier les difficultés économiques rencontrées par une entreprise qui procèdent à des licenciements économiques, je précise qu'une telle disposition figurait dans la version initiale du projet de loi travail que nous avons examiné l'année dernière et qui avait été supprimée à l'Assemblée nationale puis rétabli à l'époque par notre rapporteur, désormais ministre au Sénat, en l'absence de définition juridique du périmètre géographique, le juge français apprécie bien souvent la situation économique d'entreprises appartenant à un groupe international au niveau européen, voire mondial, ainsi que le soulignait l'étude d'impact de la loi dite El-Khomri une telle interprétation extensive pénalise l'économie française dans un contexte de concurrence mondialisée, en effet, le refus du juge de valider un licenciement économique en raison de la santé économique du groupe auquel elle appartient, mais connaît la réalité de la vie économique et est de nature à décourager les investissements dans notre pays au niveau national, des difficultés économiques cohérentes avec les règles en vigueur chez nos voisins européens apparaît donc pertinente et c'est un avis défavorable à cet amendement 196 ainsi d'ailleurs que 218 rectifier bis qui est identique pour ce qui est de l'amendement 143 rectifier 10, monsieur le président, le projet de loi travail initial prévoyait un périmètre national pour apprécier la cause économique d'un licenciement, mais face à l'opposition des syndicats, l'Assemblée nationale avait supprimé la loi travail a toutefois fait un 1er pas en objective en les critères des difficultés économiques, mais si ces critères ne sont pas exemple critique comme notre commission largement souligné l'an dernier, ils ont le mérite d'exister, il faut maintenant franchir la 2ème étape, celle du périmètre d'appréciation afin d'aligner notre législation sur la pratique observée chez la plupart de nos voisins européens, c'est donc un avis défavorable. à cet amendement 43 rectifier bis, ainsi que 232 rectifier qui étaient identique pour ce qui est de l'amendement 174 rectifier terre. consisterait constituerait un élargissement du Champ de l'habilitation, que le gouvernement nous demande de lui accorder son adoption serait donc contraire à la Constitution et l'avis de la commission ne peut être que défavorable au demeurant la sauvegarde de la compétitivité économique constitue déjà un motif de licenciement économique, comme la jurisprudence le prévoit depuis plus de 20 ans, avril 1995 2 depuis l'arrêt vidéo lors de du 5 avril 1195 la Cour de cassation a nommé et je cite que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation la notion de sauvegarde Claude à compétitivité a d'ailleurs été consacré dans le code du travail par la loi travail à l'objet de cette à une moment égorgé déjà satisfait par le droit actuel, c'est donc une demande de retrait, sinon ce serait un avis favorable le 63 rectifier. L'article 30 du projet de loi travail initial prévoyait que je cite à nouveau ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique, les difficultés économiques créé artificiellement à la seule fin de procéder à des suppressions d'emplois, fin de citation, pourra nous éclairer sur ce point et nous demandons donc l'avis du gouvernement, sur cet amendement 63 rectifier pour ce qui est du 64 édifié nous demandons aussi l'avis du gouvernement sur ce sujet,

je partage les objectifs des auteurs de l'amendement, mais je pense que la rédaction retenue empêcherait le gouvernement de prendre une ordonnance pour préciser les conditions de reclassement, c'est donc un avis du gouvernement, qui a demandé par la Commission pour le 175 rectifier terre. Si on peut comprendre l'objectif poursuivi par les auteurs de l'amendement, on peut avoir des doutes sur la portée de celui-ci, s'il s'agit d'une simple précision rédactionnelle, elle n'est pas forcément utile, je ne souhaite donc pas systématiquement pour chaque habitation rappeler les objectifs de simplification et de sécurisation juridique car je ne veux pas alourdir le texte, c'est à nous, parlementaires de vérifier si ces principes seront suivies lors de l'examen du projet de loi de ratification des ordonnances, c'est donc une demande de retrait, sinon c'est un avis défavorable de la part de la commission des affaires sociales, enfin pour le 176 rectifier c'est aussi une demande de retrait, sinon ce serait un avis défavorable pour les mêmes raisons. Merci monsieur le président, quel et dont l'avis du gouvernement sur ces amendements monsieur ministre. Merci beaucoup monsieur le président, donc débat effectivement dense, intense important sur essentiellement. Le périmètre d'appréciation le périmètre mondial, il faut quand même reconnaître qu'on est Madame Lienemann, les seuls à avoir ce type d'appréciation et et en fait. Ce périmètre mondial il est pas une prime aux délocalisations, il est une prime au non-localisation parce qu'en réalité il y a un grand nombre effectivement d'entreprises dont les, les, les, les, les sièges et les cendres de décisions peuvent parfois être située à l'étranger qui font le choix malheureusement lorsqu'ils ont la capacité de choisir entre l'Italie, l'Allemagne, la France pour localiser une nouvelle activité qui pourrait passer par une extension d'une usine en France ou à la construction d'un nouvel établissement

difficile à faire, mais le nombre d'emplois qui n'ont pas été créés en France faute et bien d'un périmètre adaptés qui permettent à ces personnes lorsque leur activité effectivement évolue de pouvoir ajuster leur outil de production parce que aujourd'hui ce qui compte, c'est bien la capacité à réagir à rebondir ajuster ses facteurs de production capital ressources humaines Technologie, hé bien à la à la vie qui est de plus en plus trépidante au contexte économique qui est de plus en plus mouvant et évolutif la ceux de de la situation actuelle et que le gouvernement effectivement sur Inter ce sujet pour que, avec les partenaires sociaux, hé bien, la discussion s'enclenche et qu'une, comment dire, une évolution soit trouvée, d'ailleurs j'ai en tête lorsque avec Jean-Marc abouti Michel Forissier, nous avions travaillé sur la loi travail dans nos auditions, j'ai repris mes notes, sachant qu'on se retrouvait ce matin, j'ai retrouvé ce que nous disait un des dirigeants de Beauchamp, qui ébauche, vous savez, un système c'est pas le capitalisme sauvage dérégulé ainsi une fondation qui avait un certain nombre de règles très dans dans l'esprit capitalisme rhénan et ébauche disait mais moi on m'a refusé d'adapter parfois outil production faute d'avoir les documents du Japon et et c'est vrai qu'on peut se poser la question de la pertinence d'avoir ce type de document dans le détail et et que du coup bien moche peut être amené à prendre de décision à l'avenir de localisation qui peut-être ne nous sont pas favorables, donc encore une fois, je crois qu'il faut pas, il faut être lucide sur la situation, ne pas être je dirais dogmatique et est arrivé à évoluer, alors c'est, c'est pourquoi je comprends que la commission des affaires sociales, dans un souci constant et de cohérence, je reprends le terme clin d'oeil que le président m'adresser souhaite d'ores et déjà inscrire dans la loi un périmètre, nous, nous pensons qu'à ce stade, compte tenu de la la méthode que nous avons choisie pour faire aboutir ses réformes ô combien importante, c'est de pouvoir continuer à discuter, que les partenaires sociaux mais par définition l'ordonnance après elle, elle mettra un niveau et donc je note d'ailleurs que dans la rédaction, issu de la commission, la commission elle-même est consciente du fait que. Le niveau auquel cas stipule, c'est-à-dire la France, hé bien elle même, elle y apporte des des amodiation puisque on parle dans la rédaction de définir d'éventuels aménagements à cette règle du périmètre national et donc du coup je comprends que finalement la commission elle-même encore des interrogations et je pense que on pourrait utilement profiter des prochains jours des prochaines semaines pour lever ces interrogations et donc je propose à la commission de se rallier à l'amendement du gouvernement puisque ça permettra, du coup, je crois, de progresser et de progresser au même rythme que les partenaires sociaux dans un esprit de Concorde qui, vous le savez, caractérise l'action du gouvernement, donc tout ça pour dire que. C'est un avis donc défavorable à l'amendement 15 rectifier bis ainsi que amendements identiques 78 rectifier bis 124 165 ainsi que ceux qui sont dans le même esprit relatifs au périmètre, c'est le 196 le 218 rectifier bis le alors s'agissant du 43 activistes Monsieur Touraine, en fait, c'est le même que celui que présente le gouvernement, donc j'ai proposé un retrait au profit de l'amendement du gouvernement on est voilà pour qu'il puisse y avoir un vote qui soit émis sur celui du gouvernement le gouvernement soutient son amendement, vous l'avez compris

la loi. Travail de la dernière. En fait, a a permis à légaliser un certain nombre de critères liés à la sauvegarde de la compétitivité qui nous semble-t-il, apporte des réponses substantielles au problème que vous avez posée, donc nous sommes qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, à ce stade et c'est pourquoi c'est une demande de retrait ou un avis défavorable, comme la commission l'a également émis vous avez ces avis défavorable répétitif mais n'espère pas que nous puissions un jour conclure sur des amendements d'ici les prochains articles

qui la oralement corriger et donc il faut bien que nous prenions en compte cette rectification qui permet au gouvernement de donner un avis favorable, c'est-à-dire que, il y a l'insertion d'un notamment devant le en termes de présentation, voilà donc je je le précise pour nos débats, donc avis favorable sur le 64 identifié le 123 oui Dominique Vatrin sur lequel d'ailleurs le le président Milan disait que, en termes de philosophie, il pouvait partager naturellement le la démarche pour compléter les propos du président Milan je voulais signaler qu'effectivement ces obligation de loyauté de sérieux d'individualisation et puis de, de, de, de chronologie précise étaient des éléments qui était

le terme employé par le gouvernement et repris par la Commission, je crois, englobe assez largement ces ces objectifs, qui sont des objectifs effectivement partagée mais nous, nous vous proposons de d'en rester à la rédaction, sur laquelle nous sommes arrivés à tomber d'accord avec la commission,

et justifiée. Réflexion volonté de, de, de sortir d'une réflexion limitée à l'échelle nationale quand il y a une multinationale alors faut le dire, hein, qu'est ce qui est dans le viseur, c'est l'arrêté de la Cour de cassation, comme l'a dit Jean-Louis Touraine qui oblige la société mère à venir au secours de sa filiale. Je dois vous dire dans ma région, mais je crois que c'est national, les investissements étrangers n'ont jamais été aussi importants en ce moment. Et la volonté, il faut le dire, d'Emmanuel Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie cette faire sauter ce verrou pour donner un impact symbolique pour attirer les investisseurs étrangers et lui qu'est-ce qui préfère, lui, préfère la vieille revendication du MEDEF. Les licenciements économiques doivent être définis par l'accord d'entreprise qui s'impose au contrat de travail. Voilà, c'est comme ça, il faut dire les choses, on est dans plein néolibéralisme sur la fragilisation ça ça se ça se traduira par une fragilisation terrible des salariés. 2ème chose le solde de derme planche mens DPS. Avec les périmètres sont proposés, ça pourrait faire baisser selon l'ensemble des syndicats de 35 pourcent l'ensemble des la dernière chance sur les reclassements allégé, il existe sur cette question une juridiction rigoureuse de la Cour de cassation qui dit tout pour l'emploi. il faut éviter les licenciements et ils faut reclasser, hé bien cette juridiction est aussi dans le collimateur des ordonnances, j'ai regardé l'amendement du gouvernement de 232 rectifier je vous dire franchement un peu donnerait le sens de cette amendement c'est noyer le poisson, pour reprendre un oxymore, on pourrait dire qu'il est d'une obscure clarté l'idée c'est de noyer le poisson et de mettre en place des ordonnances qui seront explosives et qui vont se traduire par une une fragilisation extraordinaire des salariés. Lègue Madame Lienemann pour explication de vote. J'ai bien entendu l'argumentaire de monsieur Ministre ministre qui essaie de nous expliquer que c'est en permettant de licencier et de prendre en compte uniquement les licenciements économiques sur le territoire national, donc on vous qu'on pourrait attirer les entreprises étrangères pour venir investir en France, d'abord je voudrais dire, faut arrêter de ce déclinisme ambiant. Parce que nous sommes une des Terres et plus attractive pour l'investissement privé, qui a d'ailleurs augmenté de 35 pourcent et et d'ailleurs, Madame le Ministre, qui n'est pas là aujourd'hui le sait très bien puisqu'a rapport du Business France qui explique cela qu'est-ce qui fait que les étrangers viennent en France

c'est là-dessus qu'il faut mettre la comme c'est là-dessus qu'il faut qu'on disent aux entreprises étrangères qui veulent venir son territoire national bienvenue mais il faut, il faut combattre les prédateurs, ceux qui viennent chez nous pour tirer des brevets et des marques, des profits des subventions de crédit emploi recherche pour ce pour partir, après, c'est cela qui vont combattre et c'est à cela qu'on ouvre, on fait des ponts d'or en leur permettant de se dispenser d'avoir à payer très cher et et a rendu facile les licenciements économiques dans nos entreprises françaises c'est pas la bonne stratégie pour être attractive et ça ne fait qu'accroître la fragilisation de de nos concitoyens ou 12 avant besoin de reprendre pied dans notre industrie, nous avons besoin de redonner confiance aux salariés pour venir dans l'entreprise industriel des ingénieurs de de service, mais si c'est pour être blackboulé au au moindre coup de Joseph dans la conjoncture mondiale d'une multinationale qui a décidé que, finalement, c'était plus intéressant d'aller ailleurs pour quelques bémols de de profits c'est pas là-dessus qu'on va construire la l'avenir de la France, vous ouvrez une voix, un pont d'or au haut prédateurs mais tous nos efforts pour accueillir les investissements étrangers durable d'ailleurs le gros des investissements, aujourd'hui c'est les Allemands, ce dont on nous dit toujours : ah, ils sont vachement meilleurs que nous, hé ben le gros de la veste seulement industriel et d'investissements en France, c'est l'Allemagne, les croquettes pour chien et toute une série de choses, faut pas croire, il y a peu d'industrie lourde. Si Machar collègue, la parole est à monsieur Turin. Oui, Monsieur le président, Monsieur le ministre, je voudrais dire un mot du périmètre d'appréciation des difficultés économiques et de la place de la France dans le monde et commencez par adresser mes félicitations au gouvernement, puisqu'on a eu la nouvelle quand même de la nationalisation de STX, ça veut dire que quand on a une vision élevé de la place de notre économie dans le monde, on peut prendre des décisions courageuses mais alors pourquoi en face de cette décision qui est une décision ferme et conforme à l'intérêt économique de notre pays, on a cette amendement 232 dont Martial Bourquin relevait avec justesse qu'il est confus à l'extrême, qui ménage la chèvre et le chou qui vient finalement favoriser la prédation, ça a été dit par mes collègues, monsieur le ministre parlait de d'une prime au non-localisation mais si c'est pour permettre à des prédateurs de venir chez nous acheter des entreprises prendront les brevets licenciés nos salariés puis partir à l'étranger alors effectivement ces localisations là nous n'en voulons pas si cet amendement a pour but de préparer les prochains Molex nous n'en voulons pas, donc moi je pense qu'effectivement à un moment où le débat économique mondiale est organisé autour de réflexion sur le Big Data, un débat entre l'homme ce qui que Martin Koerber sur l'Intelligence artificielle ou certains bout de la planète, prépare le véhicule autonome si notre sujet, nous c'est d'abaisser nos défenses d'organiser une forme de dumping généralisé pour plutôt favorisé le low-cost que l'investissement productif que l'investissement sur le capital humain, alors je pense qu'on n'a rien compris à l'évolution de l'économie mondiale et pour reprendre que disait Madame Bouchoux, on aimerait avoir quelques éléments qui était cette vision de l'économie en quoi ce qui est fait cette désorganisation Derek cette dérégulation cet abaissement des barrières protège nos entreprises, nos salariés notre économie nationale en rien, donc je pense qu'il faut qu'on soit ferme, le gouvernement a été capable de l'aide surexcités X, il faudrait qu'il le soit aussi sur ce périmètre d'appréciation des difficultés économiques. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, c'est finalement la 3ème année que nous discutons puisque ce débat, nous l'avons eu longuement à la fois sur le périmètre et les critères dans la loi, croissance et activité en 2015 dans la loi El-Khomri on a réglé effectivement une partie du problème en clarifiant les critères et aujourd'hui, alors moi je vais aller vite mais on discute du texte de la commission et nous avons eu une commission désaccord puisque la commission a choisi de fermer complètement le l'opportunité de discuter notamment de ce point important avec les organisations représentatives, puisque la concertation elle continue Madame la ministre, ce pas là ce matin, il n'est pas à la plage elle est effectivement attelé à sa concertation qui continue donc ce que je veux dire, donc notre position, elle est constante par rapport, le texte de la Commission, donc il faut pas voter les amendements de suppression Sion qui vont 12 à 17 ou même celui du 12 parce qu'on parle de la Commission et je propose qu'on se rallie le texte de Monsieur Touraine du groupe socialiste, c'est le même que celui du gouvernement, alors on va pas faire des préséances ici celui-là parce qu'il est, avant qu'est voté, c'est le même pas ce qu'il laisse ouvert la discussion il n'enferme pas le gouvernement dans le périmètre strictement national, c'est ça le sujet, parce que si on fait ça, ça, c'est pas la peine d'avoir des discussions avec les organisations représentatives y compris c'est une habilitation, après il y aura la ratification et j'espère que la ratification elle la discussion qu'il y a donc, si ce que je reproche à la Commission, donc je propose qu'on vote l'amendement du gouvernement ou celui de Monsieur Touraine, il n'y a pas de préséance, c'est le même. Monsieur le président Monsieur Miss monsieur plein la commission, mes chers collègues. Moi, j'ai cru en relisant un certain nombres de pages du programme de l'actuel président de la République d'un côté, on voulait libéraliser je comprends bien logique je ai pas une antilibéral farouche et d'un autre côté, on voulait sécuriser et les 2 à condition de fournir un équilibre pouvait être quelque chose d'intéressant néanmoins je constate que dans ce texte, et surtout avec la tournure prise par le travail en commission que. On libéralise à tout va et on sécurise rien et j'allais dire au contraire on déverrouille à tous les étages des obstacles imaginaires et on a, ça a été dit, dont on pense que cela va envoyer des messages subliminaux à des investisseurs internationaux. Nous pensons que ça n'est pas ainsi que cela fonctionne et je me permets de nouveau de demander au ministre lorsqu'il m'entendra, quelles sont les études d'impact qui prouve à l'international que ce que nous faisons en ce qui concerne le périmètre en ce qui concerne les échelles en ce qui concerne tout ça va parler aux investisseurs japonais ou allemands lorsqu'ils viennent en France, donc moi je pense que nous sommes en train de prendre des décisions qui sont lourdes de conséquences, c'est juste 50 ans de droit social et négociation qu'on est en train de faire passer à la trappe, pourquoi pas, je dirais que ça n'est pas une opposition de principe, mais moi ce que je demande, ce sont des preuves un certain nombres de choses tangibles qui nous montrent que c'est déverrouillage vont être porteurs d'emplois pérennes, non délocalisables parce qu'excusez-moi mes chers collègues, si on rate ce coup-là, c'est la double peine, c'est-à-dire qu'à la fois on a dérégulé totalement notre marché du travail, mais en plus, ça va être la porte ouverte, ça a été dit avec éloquence par Marie-Noëlle et d'autres collègues aux pilleurs qui vont spolier nos économies qui vont prendre nos brevets qui vont prendre nos savoir-faire et qui vont nous laisser nous nos chômeurs qui ne sont pas délocalisables, donc moi je pense que c'est un vrai problème et si je me réjouis de voir le ministre le Moine, je me faisais une joie ce matin en toute courtoisie si Madame la ministre était venu de lui poser quelques questions quant aux excellentes opération que visiblement elle est en mesure de faire connaissant fort bien le système capitalistique et évidemment quand on a des personnes qui sont aussi doués pour être capable de gagner en une journée ce que vous gagnez des milliers de smicards, je pense que nous ne vivons pas dans le même monde et je me pose vraiment la question du modèle de société que nous voulons.

et plus juste, donc, je le reconnais volontiers mais pas très opérationnel, toutes les grandes entreprises au niveau mondial peuvent déplacer. Partiellement de manière plus ou moins justifiées, la création de valeur ajoutée en fonction de la fiscalité locale, faut pas voiler face, c'est une réalité, c'est une possibilité, certaines le font légalement et dans des proportions acceptables et d'autres le font de manière éhontée mais ce n'est qu'une échelle d'un phénomène qui, je dirais qu'il est absolument incontrôlable et je dirais que c'est aussi la pratique d'entreprises françaises, y compris certaines ayant des participations de financière de l'État, c'est-à-dire à capitaux d'État, je pourrais vous citer des exemples pas le faire ici, mais un sûrement entreprises dites d'État anciennes entreprise ont cette pratique sur certaines de leurs activités, notamment lorsqu'il s'agit de flottes de véhicules d'avion ou autres qui sont possédés par une filiale, je dirais de SCI qui qui effectivement a son siège à l'étranger, moi je considère que ce n'est pas Henri défiant nos nos protections que nous empêcherons le départ de certaines entreprises, le territoire, celles qui voudront partir de toute façon, fermeront, il y aura des contentieux dure et ça ne servira à rien de faire une protection artificielle mais nous serons au contraire moins attractifs pour attirer les investissements étrangers en France et donc à mon avis, la création d'emploi parce que malgré tout, je dirais, le régime fiscal la flexibilité reste à côté de d'autres critères qui ont été cités par Madame Lienemann reste un élément de localisation des investissements étrangers dans notre dans notre pays, alors bien sûr, à l'avenir, on souhaite que le périmètre européen soit le périmètre pertinent mais ça suppose auparavant un petit peu plus harmonisation sociale et fiscale avant qu'on puisse retenir ce périmètre budget après je voudrais vous citer un exemple : si demain, Hubert à des salariés en France si Hubert perd contre l'Urssaf dans le contentieux qui qui les opposent non mais si Hubert avait des salariés puisqu'il me demande de roquettes de requalification, vous seriez amené si Hubert les licenciés apprécier le périmètre international d'Hubert il bien le périmètre international d'Hubert vous amènera à constater que si une entreprise en très grande difficulté, c'est le groupe qui est le plus endetté et qui a des résultats d'exploitation absolument catastrophique mais c'est sur un modèle totalement différent, oui, vous auriez une conclusion mondiale qui effectivement peut permettre à Hubert de licencier parce que c'est un un groupe qui est en grande difficulté, donc voilà, donc je crois qu'il faut quand même bien regarder les choses dans une économie qui n'est pas quelque chose, merci, cher collègue, je je conclu simplement en disant qu'on viendra la mi-temps de la Commission, tout en considérant la bonne foi, disons du gouvernement dans la manière dont il présente les choses. La parole est à monsieur le caddie. Pour 2 minutes 30. Et je vais revenir sur les amendements de suppression et à écouter Madame Bouchoux pendant 30 ans, on va faire des travailleurs pauvres et précaires tant, professeur d'économie, je sais pas si elle pense que dans les 30 dernières années, nous avons créé une génération de chômeurs riche en 1998 Martine Aubry déclarait qu'il valait mieux être chômeur en France que travailleur au Royaume-Uni, c'était il y a 20 ans. Le modèle de chômage de masse non sous asthme pas notre jeunesse, elle souhaite un autre avenir, les entreprises se joue des frontières pour éviter des pratiques abusives, il faut un développer une approche européenne 2 que ces pratiques soient connus du public, du grand public au Royaume-Uni, certaines pratiques fiscales d'entreprise américaine par exemple, Starbucks, qui visait à éviter de payer de l'impôt dans le pays, le Roux valu de gros dommage pour l'image de la société, c'est le client qui a affecté leur politique et leur décision, le client a beaucoup plus de force que la loi pour lutter contre les pratiques potentiellement abusives que certains dénoncent parfois avec justesse, donc nous ne voterons pas ces amendements de suppression concernant l'amendement 230 de rectifier bis du gouvernement. L'ex-prévoyance professionnelle de la ministre, ces propos votre compréhension du sujet, monsieur le ministre vous remarque pertinente vous avez siégé avec nous et vous l'avez rappelé tout ça nous incite à faire confiance au gouvernement dans sa capacité à évaluer et à appréhender la pertinence du périmètre avec pragmatisme. cependant nous partageons l'avis de la commission, vous le savez, et nous pensons que le périmètre national doit être préservé. Nous sommes convaincus que vous êtes en capacité de faire preuve de pragmatisme et vraiment nous allons devoir, hélas, ne pas voter votre amendement merci. Merci mon cher collègue, la parole comme monsieur Laménie. Oui merci monsieur le président, Monsieur le ministre, chers collègues, concernant ces 17 différents amendements et on peut aussi comprendre les inquiétudes de bon nombre de nos collègues, tous ceux qui sont présents dans cette hémicycle parce que je crois que il y a quand même des inquiétudes tout à fait légitime mais certains de nos collègues ont employé le terme prédateur, bon, je m'y associerait aussi volontiers parce que on s'aperçoit que je dirais il y a des chefs d'entreprise, honnêtes, puis d'autres qui le sont beaucoup moins con sur certainement moins de scrupules alors concernant les explications de Monsieur le Ministre, qui connaît bien aussi notre institution et nous départements également, mais dans nos départements respective, ont, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui tombent pas mal, mais d'autres aussi qui sont malheureusement aussi en difficulté, bon dans mon département aussi y aller, malheureusement des des dossiers qui sont aussi en attente au niveau du département des Ardennes et beaucoup de collègues aussi on peuvent aussi témoigner mais de l'autre côté, on s'aperçoit que ce texte essayent aussi de simplifier les choses, mais comment simplifier, quelle est la la marge de manoeuvre parce qu'on s'aperçoit aussi que bon nombre de chefs d'entreprise en particulier plutôt dans les petites entreprises Bailly il galère aussi dans les procédures dans les difficultés et tout et puis aussi bas dans l'amendement du du gouvernement que je n'ai pas trop non plus trop compris en terme de lisibilité parce qu'on parle de périmètre géographique, on parle de branches d'activité, bon c'est pas simple comment aussi parce que il y a aussi la les transpositions avec le droit européen et les contraintes par rapport à l'Europe parce que on s'aperçoit que dans notre pays, on fait pas ce qu'on veut et puis on a aussi beaucoup de comptes à rendre aussi à l'européenne et aux textos liés à l'Europe, alors donc c'est aussi il y a beaucoup d'embûches et puis on a aussi beaucoup de trop de scrute rupture parce que bon nombre de chefs d'entreprises ils savent pas trop non plus à qui s'adresser, parce qu'on vaut souvent la balle alors on, on, on sait que ce texte peut peut-être améliorer les choses, mais je pense qu'il y a aussi la tâche reste immense et c'est pour ça que, néanmoins je je je garderai aussi la confiance au ou aux collègues de la commission des affaires sociales qui ont vraiment aussi beaucoup travaillé sur ces différents amendements Jean merci. Si mon cher collègue, la parole est à monsieur Daudigny. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre mais, chers collègues, je ne voterai pas les amendements de de suppression et dans le même temps, je ne soutiens pas la position de la commission des affaires sociales, du moins de sa majorité qui fixe le périmètre aujourd'hui donc au périmètre national. Alors, le sujet est d'une grande sensibilité bien sûr qu'il existe des comportements qui sont des comportements voyous et dans le nord de la France, nous avons vécu douloureusement le traumatisme de la décision du numéro 2 de litres Moine ménagé dans le monde de déplacer à Lodz, en Pologne, une usine, qui fonctionnait parfaitement bien à Amiens, alors heureusement une solution de reprise, a pu être trouvé, mais ces comportements ne valent pas heureusement un jugement général sur l'ensemble du comportement des chefs d'entreprise alors s'agissant de la modification du périmètre d'appréciation des difficultés économiques, j'entends bien Monsieur ce que nous faisons figure d'exception en Europe, et j'entends bien aussi la volonté que vous affichez de lever le maximum de frein à l'implantation d'entreprises ou de groupes étrangers sur notre pays en même temps à clarification des critères de les 6 ans de licenciement économique que vous souhaitez ne doit pas constituer non plus la Constitution, la création d'un mode d'emploi qui pourraient être utilisées par les groupes pour contourner par divers plans comptables, un certain nombre d'obligations donc les modalités précises, par contre, je ne trouve pas d'autre mot à l'instant de tels comportements doivent être établies à cette, à ce jour il n'apparaît nécessaire de laisser au gouvernement, les marges de négociation avec les partenaires sociaux, donc je soutiendrai amendement du gouvernement qui est le même que celui qui a été présenté d'ailleurs par mon groupe et nous jugerons lors de la loi qui interviendra donc beaucoup plus tard, je pense qu'au début de l'année 2018 loi de ratification, nous jugerons du texte définitif de l'ordonnance. Oui, en fait, on discute à partir d'un présupposé qui a été dit et répété par le ministre au banc qui est que. Il y a des freins à l'investissement étranger en France et qu'il y a des emplois perdus à cause de ses freins et on enseigne de lever un de ses frères, moi je veux croire la ministre qui sera au Mans, cet après-midi et qui était mis en avant dans un article du Monde en mars dernier, le titre de l'article, c'était les investissements étrangers en France au plus haut depuis 10 ans et et on l'a cité l'Allemagne est devenue championne des implantations dans l'Hexagone, avec une production ou une progression de 35 pourcent du du nombre de projets, et la ministre elle-même disait l'année 2016 est la meilleure depuis 10 ans, je la cite, parce que probablement il y a des freins pour la création d'emplois dans notre pays mais et donc on ne peut ajuster, mais quand on la ministre elle-même, a analysé, c'était son job, avant d'être ministre, analysé que l'année 2016 était la meilleure et que les investissements depuis 10 ans, n'avait jamais été aussi haut, elle ne nous disait pas que la priorité était de de. Pour créer de l'emploi ici, par contre, on peut en perdre. On peut en perte si on lève le verrou, c'est-à-dire que certains peuvent trouver l'aubaine alors qu'ils sont implantés ici pour mettre au rouge leur société ici et délocalisée donc moi ce que je crois c'est que, encore une fois, ça a été souligné par quelques collègues vous partez d'un présupposé, vous passez par d'exigence pour aller toujours plus loin dans une dérégulation de la part d'un certain nombre de patrons, et pas tous d'ailleurs et en plus c'est tellement des présupposés et jeudi idéologique que jamais, vous nous dites : quelles sont vos évaluations parce qu'on pourrait être convaincu. vous nous sortez pas un rapport qui nous dirait voilà, avec ce blocage en France, on évalue les experts sont capables de le faire tant d'emplois. Perdu à cause d'un on a investissement d'investisseurs étrangers, par contre, tout le monde le sait que ceux qui viennent ici, et de plus en plus puisque, depuis 10 ans, il y en a plus, en plus, viennent pour la qualité de vie des transports, des infrastructures de notre recherche et ça vous le valorisait pas et vous faites le bashing qui fait que cette image de la France pour investir, merci, hé bien est dégradée. Je vais donc mettre aux voix. Les amendements 15 rectifier de 78 rectifier 124 et 165. Qui sont identiques et qui bénéficie de 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement qui est pour ces amendements. Est pour. Qui est contre.

qui font l'objet d'un avis défavorable de la commission est favorable du gouvernement puisque ce sont l'amendement du gouvernement et l'amendement présente. Et par Monsieur Touraine, qui sont identiques et j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la commission je vous rappelle je ne dire que la commission est défavorable, le gouvernement est favorable, il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement et le scrutin sera ouvert dans quelques instants.

Scrutin est clos et j'ai invité les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin numéro 136 sur les amendements identiques 43 rectifier bis et 232 rectifier Nombre de votants : 320 Nombre de suffrages exprimés 319 pour l'adoption 131 contre 188 le Sénat n'a pas adopté, nous arrivons à l'amendement 174 rectifier terre et on solliciter le retrait Madame de cet amendement, il est retiré merci ma chère collègue rectifier monsieur qui ont sollicité le retrait au profit du 64 expliquer les retirer et en ce qui concerne le 64ème quitter: êtes-vous d'accord pour rectifier Anne ajoutant notamment notamment. C'est OK, donc je le mets, on voit le 64 rectifier bis avec, par les mots, notamment en termes de présentation.

dont monsieur le ministre a souhaité que ce soit 20. Et puis soit rectifiée Anne ajoutant devant les mots en termes de présentation, notamment en termes de présentation, cela a été accepté par l'auteur de l'amendement qui est Monsieur, Gabe outils et je mets ou voir cet amendement 60 4 rectifier ainsi rectifié qui devient l'amendement 64 rectifier bis est ce clair pour tout le monde

nous arrivons à l'amendement 123 monsieur Vatrin, vous avez la parole pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, jusqu', quelques mots pour revenir sur la défense de Monsieur le Ministre, pour refuser cet amendement ces derniers jours en effet, le gouvernement des alignement par le bas, dans les ordonnances qui se fondait sur une jurisprudence trop complexe, je pense ici à la qualification non économique du licenciement d'un salarié refusant un accord collectif, donc le gouvernement retenu là en l'occurrence la juridiction la jurisprudence la moins favorable pour la codifié par ordonnance et ici à cet amendement 123 le même gouvernement se font aussi sur la jurisprudence mais pour refuser des clauses positive que le rapport auteur-a jugé tout à fait fondée et qui vise simplement à s'assurer, c'est quand même gros que les propositions de reclassements sont loyales sérieuse individualisé et réalisé dans un des délais précis, je pense que chacun tirera les comptes enseignements qu'il veut, mais pour le groupe SRC c'était pilotes confirme l'analyse générale que nous portons sur ce projet de loi, un ensemble de mesures déséquilibré qui aligne vers le bas les protections individuelles et collectives des salariés au profit des grandes.

Qui est contre. Qui s'abstient l'amendement n'est pas adopté, nous passons en devant 175 rectifier avec une demande de retrait et ainsi que le suivant : 160 ma chère collègue. Et nous arrivons à l'amendement 44 rectifié présentée par. Qui sait que présente Monsieur Touraine le 44 rectifier Madame Génisson, je n'ai pas vu la parole, ma chère collègue. Oui, merci Monsieur le le président je, nous proposons de substituer au terme conciliation le terme d'articulation qui endroit permet de dénoncer de façon écrite et détaillée des faits dont on offre de rapporter la preuve en justice, je fais référence en fait à la loi fondatrice de l'égalité professionnelle, la loi de 1983 la loi dit Yvette Roudy loi dans laquelle ce sujet de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle était une priorité et Madame Roudy insisté énormément Madame la ministre insiste énormément pourquoi on emploie ce terme qui est beaucoup plus fort et qui exprime une volonté beaucoup plus forte de réaliser cet enjeu et en citant Madame Roudy et la loi de 1983 je laisse à l'appréciation de nos collègues, surtout les bons l'état de la situation de la l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il y a encore beaucoup de travail à effectuer. Merci, ma chère collègue.

Vous avez la parole. Oui, explications de vote, je me réjouis que les avis soient favorables et au niveau de de notre groupe, on soutient tout à fait cet amendement qui a été très bien et brillamment présenté par notre collègue Catherine Génisson et ça n'est pas, je veux le dire ici, ça n'est pas un un amendement de détails et c'est important par les temps qui courent, où il y a un glissement au niveau linguistique, on emploie des mots à la place des autres et équité à la place d'égalité, ce qui n'a aucun rapport etc, parler d'articulation des temps, c'est quelque chose de très important compte on se bat pour obtenir l'égalité entre les femmes et les hommes et à un moment aussi où, dans notre société, il y a vraiment des mouvements inverses et des retours en arrière sur cette question où nous sommes toujours dans les entreprises à connaître les inégalités au niveau salarial au niveau de l'avancement à tous les niveaux, je pense que c'est extrêmement important et je me réjouis donc de cette, de cette position qui, j'espère, et de ce de cet amendement, qui gère espère sera votée à l'unanimité. Ma chère collègue dont je vais mettre aux voix l'amendement 44 rectifier avec 2 avis favorables qui est pour cette amendement. Qui est contre qui s'abstient, il est donc adopté le 45 qui et Madame Gillot, vous le présenter. Merci monsieur le président, alors le développement et l'accessibilité des nouvelles technologies impactent l'organisation de nos sociétés, les relations entre les individus, la façon dont nous appréhende on et comprenons notre environnement, le rapport à la culture, l'activité est au travail dans cette période charnière, nous devons faire en sorte que ces innovations bénéficient au plus grand nombre et participe du progrès partagé la ligne dont nous, dont nous discutons actuellement prévoit que les règles de recours aux nouvelles formes de travail le télétravail ou le travail à distance puisse être utilisés afin de mieux concilier vie professionnelle et V. weebi personnelle et familiale et dans sa présentation, Madame la ministre avait cité l'amélioration des conditions d'accès à l'emploi des personnes isolées géographiquement ou avec un handicap mon amendement vise à ce que le recours à ces nouvelles organisations de travail puisse être mieux utilisés au bénéfice de l'accès du maintien ou du retour dans l'emploi des personnes handicapées qui peuvent avoir plus que d'autres, des difficultés à surmonter chaque jour pour rejoindre leur lieu de travail quand elles ont un emploi, elle s'efforce d'en honorer les obligations au prix parfois d'une fatigabilité aggravée et handicapante à plus ou moins long terme, qui nécessitent des phases de repos, voire à une organisation du temps de travail compatibles les personnes en situation de handicap ont 3 fois moins d'opportunités d'occuper un emploi, je vous le rappelle, est 2 fois plus de risque de connaître le chômage, l'IGAS montre par ailleurs que le les taux de salariés licenciés suite à un avis d'inaptitude peut atteindre 97 pourcent dans dans certaines régions, représentant un énorme gâchis, gâchis pour l'entreprise qui perd une compétence et une forte adhésion à l'emploi gâchis pour la personne qui perd son identité sociale liée à son identité professionnelle, le télétravail peut et le travail à distance, organisation et concertation peuvent constituer une réponse pour maintenir un salarié dans un emploi adaptés, suite à un avis d'inaptitude ou offrir une organisation du travail permettant de recruter un travailleur handicapé. Mais au sein de l'entreprise bien sûr le télétravail et le travail à distance doivent être utilisés avec précaution dans le cas d'un protocole ou la vie, l'expérience des salariés seront précieux sur le plan de l'intégration du travailleur au sein de la vie de l'entreprise ainsi que du respect de ces conditions de travail matériel et et de ses horaires, la situation catastrophique de l'emploi des personnes handicapées impose d'envisager toutes les options d'étudier toutes les pistes, leur permettant d'accéder de conserver ou de retrouver un emploi, c'est pourquoi je tiens à ce que l'évocation du télétravail, du travail à distance soit bien associer à l'effort indispensable à faire pour l'emploi des personnes avec handicap. Nos chers collègues Thierry de la Commission, monsieur le président, emporte. Merci Monsieur Président parmi les 7 thèmes identifiés par les partenaires sociaux dans leur lettre d'intention commune qui a été envoyé en juin dernier à la ministre du Travail, le recours au télétravail pour les personnes nées comme handicapé n'est pas mentionné comme un accès à part entière, je pense qu'il pourrait être donc utile de donner un signal au gouvernement et aux partenaires sociaux en ce sens, même si le risque d'ouvrir la boîte de Pandore de l'énumération dans tous les cas de recours au télétravail, donc c'est un avis de sagesse très très très très positive. Et écoutez dont l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. de la Commission, c'est vrai que le gouvernement ne peut que souscrire je crois à la proposition qui est faite, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui, d'ores et déjà dans des accords sur le télétravail ont prévu des modalités particulièrement intéressante pour favoriser l'et personnes en situation d'handicap le recours à ce type de modalités d'exercice de leur travail comme Nestlé France ou Mediapost, mais essayons de généraliser cela effectivement et donc avis favorable à votre amendement de mesures. Merci monsieur le ministre, Madame Gillot pour explication de vote. et alors dans dans cette considération, je voudrais aussi qu'on soit attentif à ce qu'on ne considère pas que les enfants, les personnes avec un handicap moteur, souvent, on pense à ça, l'adaptation du lieu de travail, mais il y a aussi des personnes qui ont des problèmes neuro-développement qui ont du mal à travailler en collectivité qui doivent surmonter des problèmes de surcharge affective, et donc là le travailler dans un environnement familial bien bien adaptée peut permettre à ces personnes de donner le meilleur d'elle-même dans un une mission professionnelle et je crois que c'est absolument important là aujourd'hui 6 amendement est adopté, je crois qu'on aura fait un grand pas dans la reconnaissance des aptitudes des travailleurs avec handicap. Merci, ma chère collègue, Madame Prima. le plus grandement possible et à la fonction publique, ça serait une très très bonne idée de pouvoir l'étendre à la fonction publique assez rapidement et d'aller sur le télétravail, au-delà des expérimentations et des mises en place très timide, qui sont aujourd'hui en place dans les différentes collectivités.

à la majorité de la commission comme quoi un rapport, ça peut être utile parce que cette habilitation, elle est dans le droit fil de ce que nous avons voté dans la loi El-Khomri l'article 57 et à la, à la suite de s'rapport il y a une concertation avec les organisations représentatives, vous l'avez cité Llorens elles vont donner 5 pistes de travail et elles ont dit effectivement qu'elle voulait négocier sur tous les points et donc celui-là va être intégré à l'habilitation et donc bon j'ai un peu de suite dans les idées, et quelquefois c'est utile bravo donc demandé un rapport au gouvernement et ça produit ses effets, c'est pour ça qu'on a cette ouverture de l'habilitation pour tout ce qui concerne le télétravail. Merci, ma chère collègue, Monsieur le Président millions. Merci Monsieur Président, je suis en effet complètement d'accord avec Madame Bricq pour ça arrive, c'est un événement, c'est un événement, le, le, le seul problème, mais je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'un rapport, c'est extrêmement utile, ça peut beaucoup servir quand il est fait, le problème c'est que la plupart des rapports qui sont demandés ne sont pas faits, vous le savez très bien, et, et ceux qui sont faits, parfois, ne sont pas élus, donc le le vrai problème est là je vous, je vous rappelle, encore une fois, et Jean-Baptiste moins s'en souvient bien mais dans le cas de la loi El-Khomri y avait plus d'une trentaine de rapports qui avait été demandé, je reviendrai pas dessus, mais c'est la loi santé, donc j'avais été rapporteur il y avait 50, rapport qui avait été demandée dans le cas de la loi, c'est 50 rapport si nous avions voté la qui ont été exécutés dans la mesure où, en plus, ils ont été demandées il y a un an en arrière, entre-temps, il n'aurait pas été fait donc les rapports quand ils sont faits quand ils sont lus serve à quelque chose, uniquement dans ce cadre-là. Merci monsieur le président, donc je vais mettre aux voix Monsieur Savary, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le le le président je pense que le télétravail est

l'intégration là et qu'on doit avoir pour les personnes handicapées, c'est véritablement faire en sorte que, on les intègre dans tous nos décide positif législatif mais le télétravail, c'est vraiment une des possibilités de créer des emplois nouveaux, sur des bassins de vie, hein, et ça rejoint l'aménagement du territoire, avec le très haut débit dans tous les territoires, fixe ou mobile, et il faut continuer à se battre pour cela parce qu'on voit bien que c'est comme ça qu'on pourra sortir nos territoires les plus difficiles de de leur isolement. Simon gère collègues, je vais donc mettre aux voix la Mandement 45 titiller qui ont un avis de sagesse, plus de la commission favorable du gouvernement qui est pour cet amendement. Qui est contre cette amendement l'amendement est adopté à l'unanimité.

dans un arrêt du 31 mai 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que l'employeur ne peut unilatéralement, demander à un salarié travaillant à domicile d'exécuter sa prestation au siège de l'entreprise, une telle décision, modifiant l'organisation contractuel du travail, l'accord du salarié est ainsi requis, quand bien même son contrat de travail prévoirait une clause de mobilité, ils conviennent d'assouplir cette règle, faute de quoi les employeurs risqueront de ne pas mettre ce mode d'organisation, dès lors qu'il se relève révèle définitif. Chers collègues, quel est l'avis de la Commission, monsieur le président, porteur. Oui, la commission souhaite l'avis du gouvernement, sur certains amendements présentés par notre collègue. Qu'il y avait du gouvernement Monsieur le ministre. Alors Monsieur le Président, Madame la sénatrice, sur 177 rectifier terre malheureusement, ça va être un peu compliqué pour nous,

sur celui-là, en fait, vous évoquez à travers un arrêt de la la Cour de cassation, en fait, le cas des salariés les travailleurs à domicile et travailleurs à domicile c'est répondent un régime dérogatoire qui effectivement n'a rien à voir avec celui des travailleurs entre guillemets ordinaire mais qui ont choisi une modalité d'exécution de leur travail qui de façon partielle Leur permet de devrait dans des lieux tiers comme les évoquer, René-Paul Savary, donc en fait on est vraiment sur un sujet qui est totalement distincts et pour lequel il ne nous sommes pas qu'il faille à ce stade de bouger les équilibres et donc la Commission demander l'avis du gouvernement, c'est donc une demande de retrait, à défaut, un avis défavorable et vivement les prochains amendement que vous présenterez pour qu'on puisse y y arriver.

Nous arrivons à 3 amendements qui font l'objet d'une discussion commune et qui sont-ils, 2 amendements identiques, le 125 présentée par. Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président, depuis 2015 la progression du nombre d'intérimaires, serait de 16 pourcent,, s'approchant ainsi du record de 2007 avant la crise, une forme de travail qui voit l'incertitude d'incertitude, pardon, les lendemains 2 millions de travailleurs et de travailleuses précarisant leur travail et leur vie, c'est même un marché du travail précaire qui a explosé, faisant le bonheur d'un certain nombre d'entreprises de ce secteur cet alinéa vise à donner la possibilité de déroger par accord de branche la législation relative aux CDD à l'intérim, c'est la raison pour laquelle nous vous devez vous nous vous demandons la suppression de cet alinéa, et nous avons nous aussi fait des auditions et notamment rencontré les organisations syndicales à ce sujet, si c'est la loi qui fixe les règles du recours aux CDD à l'intérim, c'est bien pour protéger les salariés, car entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui a, qui a franchi, je pense que vous avez reconnu la la phrase de Lacordaire qui est assez cité assez célèbres : le contrat de travail est un lien de subordination que vous semblez ignorer dans ce texte, monsieur le ministre, il s'agirait d'une erreur que de penser que les employées les patrons discutent sur un pied d'égalité, et uniquement dans la bienveillance d'où notre demande de suppression de cet alinéa. Si ma chère collègue amendements identiques numéro 159 présenté par Monsieur des essais. Oui, merci Monsieur le Président, en effet, je défends le même amendement de suppression que mes camarades communistes en laissant la possibilité aux branches de déterminer les règles relatives au contrat à durée déterminée ou intérim, le gouvernement entend faciliter le recours à des contrats courts. Seulement, par définition, ces contrats courts sont précaires pour les travailleurs, l'absence de salaire garanti à l'issue du contrat de travail, a des conséquences néfastes, nous l'avons sous-souvent dit sur la vie du salarié, en effet, ces derniers ne peuvent pas se projeter dans l'avenir et donc de mener des projets à long court au quotidien leur accès au logement est compliquée en effet les propriétaires exigent quasi systématiquement plusieurs de bulletins de salaire et un contrat à durée déterminée, avant de leur louer leurs biens pareillement les banques impose une certaine stabilité des revenus pour accorder des prêts et donc de faciliter l'accès à la propriété, au-delà des conséquences matérielles le travail précaire engendre du stress du mal-être et nuit à la santé des travailleurs pour toutes ces raisons, la précarisation du monde du travail nous inquiète au plus haut point si les contrats courts peuvent être nécessaire dans certaines situations, comme les remplacements ou les pics d'activité doivent rester exceptionnelles, si l'on n'assouplit trop la possibilité de recours ouvrir aux contrats courts, c'est le CDI, pilier de notre droit du travail que l'on n'affaiblit et avec lui l'ensemble des chômeurs et travailleurs précaires, c'est pourquoi nous nous opposons. à leur facilitation au niveau de la branche et donc Monsieur le Ministre.

de dire à Madame Bricq qui va défendre évidemment le fait de s'adapter à l'économie avec des contrats courts. De lui dire que la flexi-sécurité dont nous parlons pas, faut pas s'arrêter Affleck si il faut assurer sécurité donc en même temps qu'on pourrait s'attendre de la part des gens qui veulent qu'il y a effectivement un peu plus de flexibilité, quelle est la sécurité qu'ils ont à mener pour que les précaires, puissent avoir un accès au logement pour que les précaires, puissent avoir un accès après que ces contrats courts soient sécurisés dans leur vie sociale et là vous faites simplement le contrat court vous multipliez la précarité, ça donnait un changement, alors qu'on sait qu'aujourd'hui c'est néfaste. Je vous remercie, je voudrais bien, mais c'est une mais. Merci mon cher collègue, donc quel est l'avis de la Commission sur ces 3 amendements Hama un Prima, excusez-moi, vous 2, vous avez la parole sur l'amendement 153 rectifie. Merci beaucoup Monsieur Président, j'étais étonné mais il est vrai que cet amendement n'a pas forcément tout à fait rapport avec les 2 précédents, il s'agit en fait d'un amendement que j'ai déjà déposé plusieurs fois sur lesquelles les gouvernements précédents m'avait promis de regarder et il est évident. Donc, ce dossier ne n'avance pas, il s'agit en fait des contrats à durée déterminée d'usage et notamment des ce qu'on appelle les extras dans la branche hôtels cafés restaurants, et particulièrement sur le domaine des traiteurs, c'est que ces contrats sont sont prévus notamment pour faire face à la fluctuation des de ses activités, or une jurisprudence de 2008 de la Cour de cassation a remis en cause les bases légales de cet audit dissipe dispositifs en considérant que la qualification conventionnelle de contrat d'extra dépendait de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, or la preuve du caractère par nature temporaire de l'emploi, et bien souvent impossible à démontrer parce que le recours aux extra-une une nécessité qu'il y a un besoin temporaire quand il y a des réceptions, des mariages, les traiteurs sont dans l'impossibilité d'avoir une vision très claire à plus de 15 jours quelquefois sur leur activité mais les emplois qui sont confiés aux salariés qui sont des emplois qualifiés de serveurs de maître d'hôtel ne sont naturellement pas par nature temporaire aussi faute de pouvoir apporter le preuve du caractère de par nature temporaire de l'emploi et même si l'employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles les jurisprudences requalifie la relation de travail de CDD en CDI et la relation de travail à temps partiel en temps complet, et ces décisions qui aboutissent à des condamnations de plusieurs centaines de milliers d'euros risque de conduire au dépôt de bilan, plusieurs entreprises déjà fragilisées, notamment chez les traiteurs parallèlement il y a eu un rapport de l'IGAS, ce rapport de l'IGAS a proposé de transformer ce contrat en cours, en contrat à durée déterminée successives qui sécurisent réel équilibre économique et social des secteurs concernés, à ma connaissance, et sur le rapport que j'ai lu ce rapport n'a pas auditionner les entreprises concernées et notamment le petit syndicat des traiteurs qui s'appelle le Synhorcat dans contexte cet amendement vise donc à permettre une reconnaissance dans la loi de la nature successives et temporaire des contrats d'usage et l'invite, par la même le gouvernement à se prononcer sur ce sujet et Monsieur, je vous demande vraiment de vous prononcer sur ce sujet parce que ça fait plusieurs années que cela dure et cela mais aujourd'hui des entreprises vraiment dans des difficultés majeures merci beaucoup. Merci, ma chère collègue qui, lui, dont l'avis de la Commission sur ces amendements. Merci Monsieur le Président, sur l'amendement 125 et 159, la commission a émis un avis défavorable je reviens donc je viens maintenant sur l'amendement 153 rectifier en effet par 2 arrêté en date du 23 janvier 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en exigeant désormais que le recours à des contrats à durée déterminée d'usage suisse Steve soit justifiée par des raisons objectives, c'est-à-dire par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, en pratique, il ne suffit plus que l'emploi occupé relève de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée, il faut que l'employeur souhaitant plus capable de montrer que dans chaque cas de figure, que les conditions d'emploi concrète rendent le poste temporaire mais cette exigence paraît justifiée sur le fond, la mettre en oeuvre en pratique très compliqué, vous avez raison là-dessus ce durcissement des règles entourant donc le CDD d'usage pose aux employeurs d'un certain nombre de secteurs, voudrais parler le cinéma, l'hôtellerie-restauration et les loisirs, sports, le BTP difficultés réelles qu'il faudra bien un jour levé, comme l'avait reconnu monsieur Macron en séance publique au Sénat au mois de mai 2015, il avait alors dit que ce sujet pourrait être traité dans le cas d'une loi sur le dialogue social, mais depuis, aucune décision n'a été prise, je souhaite donc comme vous demandez au gouvernement si l'ordonnance sur le CDD abordera la question des CDD d'usage et tirera les conséquences du rapport très qui éthique très critique de l'IGAS de décembre 2015, encore un rapport mais un rapport très critique de l'IGAS 2015, donc nous souhaitons évidemment la Commission avoir l'avis du gouvernement. Et monsieur le président, lequel et dont l'avis du gouvernement sur ces amendements, monsieur le ministre. purement et simplement l'alinéa 20. C'est un avis défavorable en fait la ministre d'ailleurs, a évoqué, je crois, non lors de l'article 1 le fait que les branches allaient désormais pouvoir. Travailler, avoir pour mission de travailler sur la gestion et et la qualité de l'emploi et donc justement dans ce cadre-là, de cette nouvelle mission qui qui qui qui a émergé aussi des des concertations avec les partenaires sociaux de ces derniers jours il y a très clairement il reviendra donc aux branches aussi hé bien de pouvoir adapter effectivement des curseurs sur ce type de de contrats au regard des spécificités des leur secteur d'activité, c'est toujours mieux de faire du du du sur mesure et donc je crois que c'est là un progrès et en même temps c'est c'est la branche qui sera amené à se pencher là-dessus, donc je crois que c'est vous aviez eu

on donne un avis défavorable à ces 2 amendements et pour répondre au sujet que Sophie Primas pose et pose à nouveau sustenter dire puisqu'effectivement, cela fait plusieurs années que elle se penche avec attention. Sur le la branche notamment HCR

délibérer et agir sur cette qualité de. De l'emploi et sur cette gestion de l'emploi, ça signifie que la les branches HCR ou assimilés vont pouvoir elle-même aussi porter un certain nombre de d'ajustement de, de, de, de curseurs pour prendre en compte, effectivement, les spécialistes ce secteur au-delà de cette réponse générale de principe mais mais mais quand même, c'est-à-dire que la branche vraiment pouvoir s'emparer des choses je, je suis très très allant, pour qu'on puisse ensemble continuer à regarder comment le dossier évolue justement comment la branche va s'en emparer parce que justement, hier je recevais Monsieur Eddy, le président de l'UMIH

de suivre ça dans le détail, donc si je prends cet engagement qu'on le concours suivent ensemble, c'est pas une une une clause de Style pour obtenir votre retrait, là c'est vraiment pour que on fasse ça parce que je comprends que, il y a eu quand même un certain nombre de travaux qui ont été conduits que il y a des attentes et que donc on ne peut pas se satisfaire juge de différer les 2 débats en débat et et donc, c'est en tous les cas, cet engagement de travail, je le prends, j'ai pas l'habitude de de pas le tenir voilà donc je vous demande, au bénéfice de ces explications. De bien vouloir le le retirer et et donc que l'on

Monsieur le Président, que je me sois simplement évoqué mais ce qu'on appelle les contrats courts. Pour certains d'entre vous, les contrats courts, c'est l'horreur absolue, synonyme de précarité, je crois qu'il faut, il ne faut pas que les abus qui peuvent être commises, c'est-à-dire le recours systématique, répétitif et permanent aux contrats courts de certaines entreprises disqualifie certains côtés positif de ces contrats courts, d'ailleurs, donc ces abus ont été commis dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public, le ministère de la justice et le groupe La Poste était quand même d'espèces gros spécialiste des contrats courts, avec des dizaines et des dizaines de CDD renouvelés dans le groupe La Poste, qui été largement condamnée il y a quelques années d'ailleurs par les prud'hommes. Je voudrais rectifier aussi certains éléments qui ont été données aux qui ont été tenus de manière imprécise ainsi 50 pourcent des des embauches aujourd'hui son billet en CDD, le stock de contrat de travail demeure

L'intérim et les CDD sont des moyens d'insertion dans la vie professionnelle, lorsque que vous êtes dans une entreprise que vous faites appel un CDD ou intérimaires, quand vous avez de nouveau un besoin quelque temps après, vous reprenez le même s'il a donné satisfaction et si votre besoin devient permanent, vous l'embauchez de manière définitive, donc il faut considérer l'intérim et les CDD, c'est pas toujours le cas mais comme pouvant être un moyen d'insertion dans le monde professionnel et dans dans l'entreprise, je voulais ce que j'ai indiquer à cet égard, il est bien normal que la branche est le rôle de régulateur et puis s'étendront restreindre et encadrer ces dispositifs de, de, de contrats courts qu'il faut cesser de diaboliser.

dans cet alinéa 20, il est prévu d'adapter par convention ou accord collectif de branche de dispositions Mattern de CDD ou contrat temporaire de travail, leur durée et renouvellement actuellement alors, mon collègue vient de dire qu'il y avait des embauches de 50 pourcent en en CDD, moi, les informations que j'avais, c'était 75 pourcent en en CDD dans les embauches actuellement, ce sont des faits, donc 18 mois d'embauche maximum pour le salarié, donc ce qui est très précaire alors ensuite, certains diront même pour Copains CDI bien sûr, mais si l'entreprise n'a pas la visibilité économique pour un CDI, l'employé doit être remercié conviennent donc par la branche où siègent bien sûr des représentants syndicaux de mettre en place des dispositions pour que le contrat de du contrat temporaire de travail soit plus long ça tête à tête, je voulais dire est très fréquent dans les entreprises notamment TPE-PME et donc cet article donc moi pour moi une bonne mesure à l'Avantage de l'employeur, oui, mais aussi de l'employé qui, ensuite, comme l'a dit tout à l'heure, Jean-Marc aboutit pourra peut-être retrouver un CDI, donc il faut conserver cette année 20.

Interrogé vous-même puisque vous même vous avez été partisan du revenu universel que vous avez voté avec nous ici, donc vous vous dites : il y a en tout cas personnellement, vous avez une solution par rapport au temps court par rapport au temps partiel, c'est de dire assureront un revenu minimum pour tous, ce qui permettrait effectivement d'avoir une stabilité et et permettent de justement combiner la précarité avec un revenu assuré. Mais ce n'est pas vous la position du gouvernement aujourd'hui. Et donc vous n'avez pas répondu.

J'entends bien pour l'entreprise, mais c'est mieux, même pour le 1er salarié comme l'entreprise va prendre quelqu'un sans se mouiller et on va faire un contrat court mais reconnaissez quand même qu'à l'échelle de d'une vie. d'une vie. Si enchaîné CDD les contrats courts d'ailleurs. Les contrats courts ont augmenté alors qu'il y a toujours le même nombre de contrats déterminés parce qu'ils sont de plus en plus courts. des contrats maintenant le temps d'embauche se réduit, ça veut dire qu'effectivement l'employeur comme je disais tout à l'heure, hé bien fait son marché, j'ai besoin qu'un jour je prends quelqu'un est-ce que les gens peuvent s'organiser sans avoir une vision à long terme. la, vous n'avez pas répondu à cette question pour les entreprises et il peut y avoir effectivement un intérêt à ce qu'il y a des contrats courts, mais pour les citoyens, ce n'est pas une solution, et vous n'avait pas apporté sinon monsieur le ministre, face au personnel en défendant le Revenu minimum, le revenu de base universel, vous n'avez pas apporté en tant que gouvernement, ou en tant que parlementaire en marche de réponse et nous sommes toujours dans la flexibilité et non pas assurer la sécurité aux citoyens. Oui, merci Monsieur le Président, ce ministre Monsieur le Président, rapporterait, chers collègues, je je voudrais vraiment soutenir cet amendement parce qu'il a une dimension bien plus vaste que celle qu'on est en train de lui prêter, ça se limite pas au secteur des opérations ponctuelles dans la restauration au niveau du tourisme mais ça touche aussi le secteur industriel, le secteur artisanal j'ai prendre un exemple, mes collègues élus de Franche-Comté le connaissent très bien si je prends l'exemple du monde C'est une appellation fromagère qu'on peut fabriquer réglementairement que du mois de septembre au mois de mars, ce sont des emplois qui effectivement sont très importants, parce que c'est souvent des des fabrications artisanales qui nécessite beaucoup de manoeuvres et en plus, ce sont souvent des femmes et des hommes qui, annuellement, on retrouve ce même emploi et sont très heureux de de le retrouver, je prends cette année semble là on pourrait reprendre et mon collègue a pris l'exemple des des Travaux publics, on pourrait prendre de tas d'autres exemples industriel, ça serait vraiment tourner le dos à l'emploi pour un nombre significatif de femmes et d'hommes donc ce sujet je si ce vote ma maintient cet amendement, je voterai cet amendement parce qu'il a une dimension bien plus importante, et c'est une place significative de l'emploi dans nos territoire à la fois pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes et c'est souvent une réponse sociétal, parce que, effectivement, je reprends l'exemple de ce que je on peut vivre dans certains secteurs, comme dans l'y compris dans le tourisme, ce je pense au ont remonté etc ou ce sont des emplois saisonniers, ce sont des réponses aussi, qui parfois satisfont très bien les familles. la parole est à Madame Bricq pour explication. Moi 125 et 159 parce que le 3ème, c'est un autre amendement, ils sont en discussion commune mais c'est pas la même chose, oui, oui, je voudrais dire à ceux qui prônent la suppression, il faut faire attention je reprends une partie de l'argumentation de Monsieur le ministre, ce travail va être confié aux branches et les branches elles sont quand même capables, elle sera organisée aussi par secteur d'activité, de, de prendre en compte la diversité de notre tissu économique, et donc il y a des il en général dans l'industrie, sauf quelques secteurs, je pense à la mécanique à la construction navale au bâtiment bien sûr puisque c'est là où on a fait les les contrats de chantier, ils ont besoin à la fois pour satisfaire à des commandes à la fois de l'intérim et à la fois d'une main-d'oeuvre qualifiée, aussi pour des durées qui peuvent être de 2, 3, voire 5 ans quand il y a des commandes forte et miss a cité l'exemple d'STX s'ils avaient pas ce cette souplesse, ils auraient pas eu certaines commandes et je crois qu'à Saint-Nazaire et sont plutôt contents quand même d'avoir des carnets de commandes pleins pour quelques années donc les branches sont quand même capables d'apprécier s'il y a, il y a des secteurs j'ai parlé de la chimie, la chimie, ça les intéresse pas trop les voilà ils ils préfèrent avoir une manoeuvre au long cours, bon je cite ces exemples, je pourrais en citer d'autres, donc je crois que le fait que les branches soit en capacité de faire des propositions à ce sujet, c'est quand même un progrès, ça donne une visibilité globale et en même temps ça apporte une certaine sécurité parce que vous avez tout le temps, dit l'année dernière, c'est la branche et la branche c'est pas l'entreprise, bon là effectivement les branches s'intéressent à ce sujet, c'est quand même un fait nouveau par rapport au début de la discussion parce que c'est arrivé hier et puis je veux dire à monsieur de César, qui m'a interpellé comme le gouvernement, j'ai dit dans mon intervention en DG que le véritable élément de sécurité professionnelle, c'était le volet que je souhaite, en haut de la Jeanne Arc du du gouvernement de la formation professionnelle et de l'élévation des compétences des compétences des travailleurs en France, ça c'est un vrai sujet de compétiton. Si ma chère collègue, la parole est à monsieur Bourquin, explications de vote. Sur la la volonté de d'augmenter encore cette précarité Daniel Gremillet, donner un exemple, je connais bien le monde, or je vous conseille, c'est un excellent fromage avec le comté sont excellents. Daniel. Sur cette question, l'avancée la plus importante a été l'annualisation du temps de travail et des entreprises, plusieurs entreprises du Haut-Doubs qui fabrique ce fromage mais aussi d'autres charcuteries, on fait en sorte qu'en hiver, où il y a la forte demande et en été, on n'est pas les mêmes horaires, c'est une première réponse et l'annualisation du temps de travail a été une réponse, en plus, nous, nous ne nous cachons pas les il faut pas se cacher, hein, je vous le dis franchement il y a l'appel à l'intérim qui est massif, l'appel à l'intérim et massif et ce que je vais vous dire chers collègues, c'est le débat qu'on va voir, on ne peut pas toujours demandés aux mêmes de faire des efforts de subir la précarité c'est terrible pour certaines personnes. Moi, j'ai, je vois des gens, des personnes qui ont 40 ans, 45 ans, qui ont besoin encore pour avoir un prêt pour avoir un appartement d'avoir la condition des parents, ça se passe comme ça la vie avec la précarité, sachez bien quand on voit des choses comme ça, ce sont des drames humains et l'explosion de la précarité pose, y compris des vrais problèmes aux entreprises, si bien que certaines se mettent à réfléchir en disant on est allé trop loin dans la précarité et et voyez, après ça, on leur dit depuis un an, vu la production, il faut des CDI, il commence à y réfléchir. Avec Intel bénéfice cette année, il faut des CDI alors sachez quand même chère collègue comme au Mans, on va voter ça que 35 milliards ont été versés aux actionnaires au 1er semestre. De cette année, la France est championne d'Europe 1 il faut le savoir, un versement aux actionnaires, championne d'Europe. Et je voudrais dire, mais bon, c'est pas une attaque personnelle, quand on gagne 1 millions 3 d'euros en une journée

Cher collègue. La parole est à monsieur Savary. Pour explication de vote. Merci, moi je demande effectivement à monsieur le ministre, de prendre en compte l'amendement de, de,

toutes mes excuses pour mon impertinence simplement j'en reviens au texte c'est vraiment ce sont vraiment des emplois locaux non d'école délocalisable effectivement qui touche des personnes en difficulté et là c'est un peu le président du dépôt d'un département qui reprend un peu la main où on est confronté avec l'insertion, les bénéficiaires du RSA qui sont touchés, justement, à travers ce ce type éventuellement le contrat d'usage pour un certain nombre de. De, de, de, d'complémentaires, entre 2 avec sauf que c'est qu'à chaque fois tenu de la truction trimestriel du RSA, on remet en cause le montant de l'allocation de de solidarité qui a versé en plus du revenu du travail, puisque c'est une allocation de subi annuités dont le calcul est variable en conséquence Monsieur Ministre ça permet à travers la reconnaissance de ces contrats d'usage. De faire en sorte d'avoir une action innovante dans le domaine de l'insertion, au-delà simplement de la politique de l'emploi pour remettre le pied à l'étrier, un certain nombre de personnes, je pense que là, on vous offre une opportunité extraordinaire de prendre en compte les les difficultés des bassins d'emploi à travers les contrats d'usage, c'est pour ça que je demandais à ma collègue de surtout ne pas retirer cet et nous pourrions le soutenir largement et ce serait vraiment la marque du d'une avancée qui va dans le sens de ce que vous souhaitez faire sur le plan gouvernemental, nous sommes vraiment des gens constructif. Merci mon cher collègue, Monsieur le Ministre, vous souhaitez intervenir. Merci beaucoup monsieur le président, dans la loin de moi le le souhait de vouloir allonger les débats, mais quand même un certain nombre de d'interrogations de remarques, suggestions. Ont été faites. Alors j'ai pas laisser accroire l'idée que, il y aurait ici les méchants qui veulent absolument pris. que justement le projet présidentiel sur lequel Emmanuel Macron a été élu, c'est un projet qui a au coeur les mobilités hé oui et la mobilité sociale aussi en 1er lieu: faire en sorte qu'on soit pas assignée à résidence, effectivement, dans des emplois précaires et donc de ce point de vue là, le gouvernement fait le choix de mettre le paquet sur la formation professionnelle, il y a un plan de 50 milliards d'euros, dont je crois 15 de mémoire qui vont aller sur ces sujets-là, et donc c'est un effort effectivement sans commune mesure sans précédent, mais parce que on a besoin aussi de nous simplement de d'enrichir nos ressources humaines, il n'est de richesse que d'hommes, disait Jean Bodin et donc on y croit, on y croit fermement et et donc d'ailleurs un certain nombre de mesures qui sont prises dans ce projet de loi, elle vise à favoriser le recours aux CDI lorsque des mesures sont prises sur les barèmes sur la sécurisation, effectivement d'un certain nombre de de modalités dans les procédures de licenciement, c'est pour que des employeurs

et industrialiser le recours à des formes de contrats qui sont effectivement courte maintenant il existe des secteurs dans lesquels par la spécificité. C'est

le sujet sur l'amendement de, de, de Sophie Primas. René-Paul Savary et et. J'entends son assistance au regard des enjeux pour le secteur tourisme mais pas que Daniel Gremillet évoqué d'autres secteurs qui peuvent être concernés, mais franchement

selon ce que la branche va pour va va faire parce qu'on côtoie la branche de pouvoir prendre la main aussi donc la branche d'elle-même, va peut-être faire des choses mais il y a pas que cette banque chaque est concerné, je l'entends, moi ce que je souhaite vraiment, c'est que on puisse y travailler ensemble, on a une clause de rendez-vous qui est pas trop lointaine, puisqu'il va venir après un projet de loi un 2ème projet de loi sur formation professionnelle apprentissage de contrat, bref, donc on a une clause de rendez-vous et là, je comprends que si on débouche pas vous soyez fondé à. Dire ben attendez voilà Là encore une fois moi de de notre souhait de prendre en compte le sujet que vous posez, dans la mesure où encore une fois, il y a eu des, des, des engagements forts en termes de cap qu'ont été posées hier après-ministre en termes de méthode voilà 16 ans celle que que je vous propose, en toute bonne foi puisque vous faisiez référence à quelques métaphores. Merci.

que je lui fais totalement confiance, je lui fais totalement confiance, comme j'ai fait confiance auparavant un certain monsieur Macron qui aujourd'hui est aux destinées de notre pays et donc je vous fais confiance et je trouve que cet amendement vous permet justement de travailler tout à fait librement puisqu'en fait il est très léger, il dit simplement qu'on permet l'accès à ces contrats dans cette certains secteurs d'activité ou les contrats d'usage sont par nature successifs et temporaire, ça fait juste couvrir donc vous pourrez vous serez pas prisonnier, vous pourrez mener vos négociations avec les différents syndicats avec les différentes fédérations, ça ne fait qu'ouvrir les possibilités du Champ de votre négociation dont je vous fais entièrement confiance comme je le faisais au précédent au gouvernement, et particulièrement au au ministre, monsieur Macron, mais je voudrais vraiment passé cet amendement pour m'assurer que ce ce cette problématique sera bien traité, je voudrais juste dire à monsieur de 16 2 et de César 2, pardon, excusez-moi, décidément, Jean bafouille, qu'il y a des contreparties sur cette sur ces contrats temporaires et ses contreparties, elles, elles prennent en fait le l'objet d'un d'un système d'assurance chômage qui est très proche de celui des intermittents du spectacle, donc il y a une contrepartie, en réalité, sur ces contrats d'usage qui est assez important, compte tenu de la flexibilité qui a demandé à ses employées au président de la commission de de regarder avec attention le rapport de l'IGAS sur ce sujet parce que le rapport de l'IGAS sur ce sujet, il pointe notamment le déséquilibre des comptes sociaux concernant ces contrats-là, ce qui n'est pas pas tout à fait le le la problématique que je pointe claquer une 1er d'usage de ces contrats par les entreprises et d'utilité de ces contrats par ces entreprises, s'il y a des déficits sociaux les régler autrement avec cette problématique, mais c'est pas l'objet de mon amendement donc pardon à monsieur le ministre je ne retire pas cet amendement parce que je veux que ce Merci, ma chère collègue de la parole de monsieur Vatrin, explications de vote. Oui, j'ai aussi pour répondre à l'argument que j'ai entendu ici 2 fois, suggérant que nous serions un petit peu en contradiction puisque, effectivement, dans le cadre des débats des débats sur la loi El-Khomri nous avons à maintes reprises le confirme : valoriser le rôle de la branche et défi et et rappeler son rôle de régulation, je crois que ce ce rôle de régulation, il est réclamée aussi par les petits entrepreneurs et s'est exprimée largement au moment de ces débats puisque sinon, si on laisse toute latitude aux petites entreprises, cela conduit à des possibilités de dumping social c'est d'ailleurs encore aujourd'hui la position de l'UdeS qui regroupe les employeurs de l'économie sociale et sort et solidaire et qui s'inquiètent d'ailleurs du texte des ordonnances et de ses répercussions en termes de dumping social dans des secteurs tels que le sport, l'animation ou l'aide à domicile. Mais ici, on n'est pas dans ce cas de figure d'un rapport branches et entreprises, on est dans le cadre de la l'encadrement des CDD que : qui est qui existent déjà aujourd'hui par la loi. Et que vous voulez transférer aux branches, hé bien moi je considère quand même que là on a un sujet d'ordre public, parce que vous l'avez dit pourcent des des embauches aujourd'hui se font en CDD, c'est intolérable par rapport aux questions de précarité que ça entraîne pour les salariés et je crois que c'est un faux argument, de dire qu'il faudrait que confie à la branche pour que chaque secteur d'activité adapte parce que les règles nationales définit bien des cas tels que de recours aux CDD, tels que le surcroît d'activité, tels que le remplacement de salariés absents ou encore d'autres situations qui sont prévues dans la loi et donc je vois pas qu'est-ce quelle souplesse supplémentaire, il faudrait encore rajouter sauf à augmenter précisément la précarité des salariés sans rien régler au problèmes économiques qui, pour qui s'peuvent se poser. Merci mon cher collègue,

les amendements identiques 125 et 159 qui ont 2 avis défavorables qui est pour ces amendements. Qui est contre. Qui s'abstient, ils ne sont pas adoptées, m'alors, nous passons à l'amendement 153 rectifier. Avec l'avis du gouvernement demandées par la Commission, c'est donc un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour cet amendement.

Il n'est pas adoptée. Nous passons à cet amendement qui font l'objet d'une discussion commune : l'amendement 51 rectifié présenté par Monsieur Touraine. Monsieur le président, Monsieur le ministre.

Il s'agit des contrats à durée indéterminée, sur une durée déterminée. Ainsi, en France, plus de 3 millions de personnes travaillent avec un contrat précaire cette précarité n'a cessé d'augmenter, passant de 4 à 15 pourcent moins moins de 20 ans, il semble donc que le développement de cette forme d'emploi ne soit pas sérieusement entravée, faut-il dans ces conditions, créer un nouveau contrat, fusse en l'appelant CDI alors qu'il sera par définition à durée déterminée non en terme de calendrier, mais en terme de durée d'un chantier ou d'une opération, c'est déjà un abus de langage s'adresse-t-on ici à notre Intelligence pour le dire avec autant d'délicatesse dans un interview accordée à la presse la ministre du Travail, avait indiqué que l'ACDI reste le il est surtout vrai qu'un CDI ne pouvait être requalifiée par un juge en CDI, puisqu'il ne saurait déjà, c'est tout à fait astucieux pour limiter encore à la fois, encore une et de quelles normes parle-t-on ici, quelle serait l'encadrement de ce contrat de chantier, il y aurait-il une durée plancher une durée plafond par exemple, seraient-ils réservés à certains secteurs à certaines classifications était en train de nous faire comprendre le moins brutalement possible que le vrai CDI doit disparaître au profit d'une d'une précarité généralisée et de ce et que ceux qui auront à contrat précaire de plus de 2 ans seront les mieux lotis : en 2009. Le ministre du Travail de l'époque voulait déjà étendre à d'autres secteurs que le BTP, les contraintes chantier en 2013, le MEDEF avait proposé un CDI de projet de 9 mois minimum et cette mesure avait été retiré au dernier moment, à la demande des syndicats, nous ne sommes donc pas étonné de le voir réapparaître aujourd'hui, nous espérons qu'il n'est pas le marqueur d'un nouveau et terrible monde et nous sommes et nous y sommes donc totalement opposé. Pierre collègues l'amendement 100 même si Monsieur Vatrin, vous avez la parole. Oui, dans le même esprit que l'amendement précédentes puisque nous visons à supprimer la la ligne A 21 de cet article, nous avons d'ailleurs toujours ici défendu les contraintes Durée indéterminée qui sont une protection pour les salariés, je crois qu'il y a pas besoin : trop de s'étendre là-dessus et que effectivement c'était mes Linia à des légitime en quelque sorte avec les contrats de chantier qui s'appelleront demain, contrat de mission, peu importe, je crois que tout simplement, le gouvernement s'inscrit dans une dynamique de flexibilisation du CDI alors on comprend bien, puisque, il nous a déjà indiqué que pour lui c'est l'insécurité des salariés qui crée le dynamisme économique, nous avons montré que tout cela part d'un postulat tout à fait et René qui a montré que des échecs depuis 30 ans et qui comme méconnaît profondément le caractère nécessaire d'un CDI aujourd'hui et c'est bien cela qui est important de prendre en compte parce que comment voulez vous louez un appartement, comment voulez-vous contracter un emprunt ou à effectuer un achat d'importance si vous n'avait pas un CDI, le CDI aujourd'hui bah, c'est un constat, c'est une condition signer quoi, non pour s'installer dans la vie et pour avoir une vie digne de ce nom. Et si vous en doutez, et je vous demande véritablement d'aller demander à tous ceux qui aujourd'hui ont un contrat CDI intérim ce qu'on leur rétorque lorsqu'ils vont chercher un crédit lorsqu'ils veulent trouver un logement, leur dit : ah mais non, il y a le mot intérim.

refuser tout pareil leur demande parce que il y aura CDI chantier parce que il y aura CDI mission et donc le problème, à notre avis, c'est de régler le problème de la non application des règles qui limitent le recours aux CDD, beaucoup d'entreprises ont été condamnés, j'en ai cité des exemples déjà par le passé et ni la situation actuelle n'est acceptable ni ce que vous nous proposez qui ne ferait que l'aggraver.

avec le présent projet de loi, le gouvernement entend développer les contrats Durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération les femmes. C'est des projets durée interne de durée indéterminée n'apparaît que dans le nom de ce contrat qui sonnent aux oreilles comme un étrange oxymore,

autrement dit, ces salariés vont tout de même subir la précarité engendrée par les contrats de travail à durée déterminée et les conséquences néfastes qui les accompagnent, je ne reviendrai pas sur les difficultés rencontrées par ces mêmes salariés tant sur le plan matériel que sur le plan physique le gouvernement prétend que cette appellation permettra aux salariés d'être plus facilement, titulaire d'un bail ou de bénéficier d'un prêt seulement la simple lecture du contrat montrera l'artifice du dispositif, en plus de cela, ces salariés ne vont à ma connaissance, mais peut-être aurons-nous des précisions ne vont pas bénéficier des rares avantages que procurent les contrats courts, à savoir la date précise de la fin de contrat pour mieux l'anticiper, éventuellement, préparer un autre travail oui le versement de la prime de précarité, on le comprend bien, c'est donc sous cet artifice, la double peine pour les salariés titulaires de ces contrats à durée d'était indéterminée pour la durée d'un chantier, une opération. Car collègues l'amendement 215 rectifier bis qui c'est qui le présente monsieur Assouline. Oui, c'est un c'est un amendement de de repli, bien entendu, puisque je je tiens l'amendement présenté par Monsieur Touraine, qui propose la suppression donc je plaide d'abord pour la suppression pour qu'on comprenne bien, et là encore l'inventons pas des histoires qui a demandé ça. Le MEDEF 2013, 2015, il est revenu à la charge, ça ne vient aucunement du monde du travail puisque vous dites que c'est pour le bien du monde du travail, faut quand même remarquer pendules à l'heure. Donc ça ne vient pas du monde du travail ensuite, j'ai l'impression que ce contrat qui effectivement montré des fois tout le cynisme qu'on peut avoir dans la politique, il y en a pas mal, mais aussi pour un certain nombre de hauts fonctionnaires pour habiller les choses parce que franchement. C'est un contrat à durée déterminée, y compris moins bien protégés cumule les désavantages et de l'intérim et du contrat à durée déterminée, mais parce qu'on l'a appelé : contrat à durée indéterminée, on pense qu'on a réglé le problème, enfin il y a pas un salarié, lui qui est dupe sauf que voilà, c'est une façon d'habiller, on fait du mal, on est gentil, bon ça ça à force ça va irriter beaucoup, notamment ceux qui vont être frappés par cela, en plus, nous voyons qu'il y a une une précarité déjà très forte des secteurs où se concentre la précarité et ça va l'accroître parce que ailleurs, comme certains l'a souligné, la chimie et d'autres secteurs, on embauche à durée indéterminée, ça changera rien et d'ailleurs, je le disais hier une expérience pas une expérimentation d'ailleurs une oui on peut parler d'expérimentation mais en Hollande, ils ont aux Pays-Bas, ils ont fait ça. Avec l'argumentation que ça va créer de la souplesse, et donc de l'embauche et ils ont constaté que ça n'a pas embauché, mais par contre qu'à l'intérieur des entreprises, ça crée une fragilisation et et ça des personnels déjà fragilisé et ils sont en train, c'est ce que disait le monde hier de prévoir d'arrêter avec ça et de revenir à l'ancien système, avec quelque chose de clair indéterminée déterminé donc ce que j'ai proposé, c'est un moment de repli pour l'expérimenter merci Gilles à la suppression ne passe pas dans le secteur du numérique et des Start-Up et d'évaluer à merci gère les bons effets. La parole est à la banque demande 19 à rectifier bise Monsieur Savary vous le présenter. Merci, oui ça va dans le même sens, de propositions d'ouverture à des contrats, je vous propose le contrat de croissance : voilà le contrat de croissance, n'est que la décroissance. Par cet amendement, donc il s'agit de créer ce contrat de croissance, un contrat à durée indéterminée qui serait basé sur des objectifs collectifs liés à des indicateurs économiques prédéterminé, qu'il conviendra d'avoir atteint au terme d'une période définie, en effet, il serait tenu compte dans le contrat de travail de ses objectifs, tels que le développement des parts de marché, le lancement d'une nouvelle activité, d'un nouveau produit ou d'un nouveau service l'atteinte de ces objectifs impliquerait automatiquement la poursuite du contrat de manière indéterminée, en revanche, le fait que ces objectifs ne soit pas atteints constituerait au terme de la période définie d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le contrat de croissance se différencier du contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération dans la mesure où il aurait vocation à ne pas avoir de termes excepté si les objectifs collectifs liés aux indicateurs économiques prédéterminé ne serait pas atteint le contrat de croissance sera alors un contrat visant à favoriser les emplois pérennes. Merci monsieur le président, le projet de loi restreint la possibilité de conclure des contrats de mission à l'adoption d'un accord de branche, les entreprises ayant besoin de recourir à ce type de contrat risque donc d'être bloquée si la branche de leur secteur professionnel n'a pas encore conclu de convention ou d'accord afin de résoudre cette difficulté, le présent amendement propose qu'un accord de branche qui aurait été conclu sur cette question au niveau professionnel ou interprofessionnel dans un autre secteur puisse être élargie au secteur professeur professionnel ou à la branche d'activité concernés 206 heures suivant oui et donc cet amendement de même nature propose qu'à défaut d'accord de branche conclu dans un délai de 12 mois à compter de la publication de la future loi d'habilitation, les contrats de mission puisse être mises en place dans le secteur considéré. Chers collègues, quelle avec la Commission sur ces amendements, Monsieur le Président, rapporteur. Merci Monsieur le Président l'amendement 51 rectifier bis, les partenaires sociaux semblent souhaiter donner le monopole aux accords de branche en matière de gestion et de qualité de l'emploi, ce faisant, les accords de branche fixerait les règles du recours aux CDD au contrat d'intérim et aux contrats chantiers dans les entreprises relevant de la branche je partage cette analyse, qui permettrait de fixer un socle de règles communes pour éviter la concurrence sociale déloyale entre entreprises, c'est dans cet esprit que la commission d'affaires sociales a souhaité préciser que le recours aux CDI chantier devra respecter un cadre commun fixé par la loi qui distinguera ce qui relève de l'ordre public absolue déjà de branches des dispositions supplétives c'est donc pour cet amendement 51

: le 1er c'est qu'il écrase l'encadrement des accords de branche, auquel le gouvernement et les partenaires sociaux et le Sénat sont attachés, la seconde est que la notion d'expérimentation mentionné dans l'objet n'apparaît pas dans le dispositif, c'est donc une demande de retrait, sinon ce serait un avis défavorable pour le 19 rectifier bis, la notion de projets de croissance, mon cher collègue séduisante sur le plan intellectuel n'a pas d'existence juridique, elle apparaît donc compromise dans la notion d'opération qui est bien plus large que celle de projets de croissance listant les projets de développement de l'activité d'entreprise de l'emploi, comment identifier de tels projets, le plus simple, selon moi, est justement de faire confiance aux partenaires sociaux de la branche pour définir les conditions de recours au CDD branches comme le prévoit l'habilitation le législateur ne peut pas prévoir a priori et abstraitement tous les cas de figure autorisant utilisation de celle des chantiers, ce serait donc un retrait ou un avis défavorable pour le 205 rectifier le présent amendement ainsi d'ailleurs que, suivant le 206 précise le sens des mesures que le gouvernement était habilité à prendre pour favoriser et sécuriser le recours aux contrats chantier il vise à ce que, en l'absence d'accords de branche, les entreprises puissent avoir recours à des contrats chantier sur la base d'un accord collectif conclu dans un dans une autre branche et élargie par une décision du ministre du Travail de remarques sur le sujet,

Je voudrais souligner que l'élargissement n'a de sens que si la branche d'accueil à des caractéristiques sociales et économiques proche de celle de la branche d'origine, par exemple, un accord devra en Chine dans le de plasturgie pourrait être élargie à la branche de l'imprimerie, mais pas à celle des architectes donc la Commission s'en remet à la sagesse plutôt négative du Sénat sur le sujet 206 rectifier c'est une demande de retrait, sinon ce serait un avis défavorable. Si Monsieur le Président, quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président sur avant de donner un avis, amendement par amendement quelques précisions naturellement sur la position du gouvernement sur ces contrats de chantier s'est dite chantier il faut voir de quoi on parle en terme de nombres 20000 salariés. Sur 23 millions de salariés 1 pour 1000 1000 1 pour 1000 voilà, non mais c'est important de savoir, voilà de quoi on parle, parce que très clairement

l'idée. Elle est quand même d'offrir de la visibilité tant pour le salarié qui employeur la visibilité, c'est que le salarié, il va pas enchaîner des CDD de 6 mois, ça va être par exemple pour l'arrestation d'une tâche qui peut prendre de 3 ans, 4 ans et à telle enseigne que on parle beaucoup de STX aujourd'hui et le gouvernement sera amené à s'exprimer, je crois, dans l'après-midi, sur ce sujet-là, mais si on prend l'historique de de de STX, à un moment, les partenaires sociaux. Employeurs comme salariés, ils étaient arrivés à un accord assez novateur impact territorial, justement, dans lequel il y avait en terme de ressources humaines, le recours pour un certain nombre de chômeurs de personnes en recherche d'emploi, à un CDI chantier accompagnés de dispositifs de formation professionnelle accompagné parce qu'effectivement, il faut pouvoir prévoir aussi, à l'issue du chantier, la possibilité pour ces personnes de continuer sur d'autres missions sur d'autres emplois, quelle qu'en soit la forme tout ça pour dire que malheureusement ce pacte territorial qui avait été élaboré avec les partenaires sociaux, il n'a pas pu voir le jour, justement puisqu'il a buté sur l'absence de dispositions législatives permettant de sécuriser untel accord c'est pourquoi vous nous voyez aujourd'hui gouvernement prévoir dans le ce texte habilitation une mention par rapport à notre souhait de favoriser sécuriser ce type de dispositif et je crois qu'on est, voilà, donc je voulais vraiment rappeler ces ces, ces, ces principes rappelés également le nombre de personnes concernées, rappeler la dimension vertueuse, on voulait donner lorsque les partenaires sociaux s'en occupait il y avait le souci constant des uns et des autres, Guillemette de la formation aussi, bref, on le sait, on peut plus sous la toise. Y 2. Du CDI de 40 ans dans la même entreprise ce monde a changé et et ce serait vain que de vouloir commettre des lignes Maginot totalement illusoire, là encore il s'agit pas de précariser, il s'agit au contraire de trouver des modalités d'organisation qui permettent à des salariés de revenir afin de revenir à l'emploi parce que, en en l'occurrence il jette chômeur et donc je crois qu'il ne faut faire de mauvais procès au gouvernement suisse sur ce sujet-là et pour terminer, par exemple avec le sujet de la construction navale, lorsque ce type de dispositif n'ait pas pu être mis en place il y parfois sont des formes d'emploi qui étaient encore moins sécurisées ont été, du coup, la mise en place, donc c'est pour ça que je crois que. Parfois, il faut vraiment là-dessus avoir un regard je crois très dépassionnée et c'est donc le la raison pour laquelle. Sur les amendements de suppression sèche de La Linea 21 donc le 51 rectifier bis, le 126 le 164 donc, ce sont tous des avis défavorables, tout comme la Commission, et ensuite sur l'amendement 215 rectifier bis de monsieur Assouline qui prévoit une expérimentation effectivement dans le secteur du numérique qui peut le plus peut le moins et je comprends que pour vous, qui peut le moins et mieux, mais nous on souhaite garder l'épurer et faire en sorte que, il y a pas de restrictions, un seul, un domaine, un avis défavorable pour le gouvernement sur l'amendement 19 rectifier bis de monsieur présenté par René-Paul Savary qui, malgré tous ses efforts, n'a pas pu convaincre la Commission et le gouvernement non plus sur le caractère juridique de cette notion de projet de croissance, on pense surtout je sénateurs que la rédaction actuelle permet en réalité de couvrir des oui, des opérations de croissance, donc, c'est donc un avis,

pour lequel. En fait, les auteurs de l'amendement propose de prévoir d'ores et déjà l'échec d'un accord de branche sur le fait qu'il n'est pas d'accord, qu'il soit atteint dans une branche hein sur ce sujet-là, en fait, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement d'en rester au droit commun, parce que le droit commun prévoit d'ores et déjà ce qui peut. Devenir survenir dès lors que, une négociation n'aboutit pas dans une branche rien n'interdirait donc un d'appliquer les dispositions du 22 61 17 du code du travail au contrat de chantier et si une carence et constaté le ministre du Travail peut d'ores et déjà procédé à cette extension et donc l'affirmer dans le projet de loi d'habilitation serait redondant et j'ai entendu sur ces bancs, le souhait de simplification, le souhait d'une. Pas alourdir de façon excessive des pages d'un. Déjà très fourni et donc je vous propose, par cohérence, hé bien de de retirer cet amendement à défaut sera ma vie défavorable

Nous voterons contre ces amendements mais je voudrais en profiter pour rappeler un peu l'histoire parlementaire alors on l'appelle contrat de mission contraint de chantier bon verra l'appellation qui sortira du travail qui est confiée aux branches, peu importe le non mais il y a un nom légal, il s'appelle le contrat à durée déterminée à objet défini et il y a été intégré son principe avec une expérimentation qui a duré 5 ans dans la loi de du 25 juin 2008, donc on ne découvre pas ça à la faveur de cette habilitation et il a été vu le principe et l'expérimentation à la durée, 5 plus 5 ans puisque c'est en 2014, que nous avons eu à examiner une loi relative à la simplification de la vie des entreprises qui était présenté à l'époque par Thierry Mandon qui était en charge du sujet de la simplification et c'est la loi du 20 décembre 2014 mal défini vraiment après cette expérimentation les règles de ce contrat et, pour faire vite, c'est un contrat limité à 36 mois etc etc je ne décrète pas mais ce que je veux dire c'est que ici on parle de contrat de chantier parce que et de contrats de mission, je n'y reviens pas, j'ai déjà dit ce que j'en pensais du bien et pour l'économie pour l'emploi et pour les salariés comme pour les entreprises qui donne une souplesse et une sécurité en même temps, mais ce que je veux dire c'est que il a été beaucoup utilisée aussi à la suite de la loi de 2014 pour des des ingénieurs et des cadres, et notamment dans ce qu'on appelle l'industrie du futur, il a été, c'est très utile pour faire appel à des cadres, souvent de haut niveau, des ingénieurs pour trouver des nouveaux process qui vont accélérer la compétitivité de notre industrie en France, donc je pense qu'il faut faire très attention et le confier aux branches qui connaissent leur secteur d'activité, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, ne non pas dans la pharmacie, Madame Lienemann, c'est surtout dans un dans des industries de haute technologie de pointe, donc ce n'est pas forcément la la pharmacie je crois pas en plus mais est-ce que je veux dire c'est que, pour terminer, monsieur le président, il faut effectivement le confier aux branches parce que c'est elle qui vont définir dans quel secteur d'activité,

Oui, je crois qu'après que tout ce que nous avons entendu sonner ça mérite quelques précisions et quelques rectifications. Alors je ne doute pas que le l'ambition aller d'un tendre 90 pourcent de de CDI, vous ne l'accompagner avec ce système-là, vous allez-y arriver était vite, je suis persuadé que ça aura beaucoup de succès, je ne doute absolument pas du succès que ça aura auprès des entreprises, et vous pourrez ensuite en terme de statistiques vous glorifier d'avoir mis en place un système qui fonctionne le problème et je vais essayer d'être aussi clair que possible, c'est la généralisation du CD Chantier à la place du véritable CDI CDI c'est pas le fait de transformer des CDD en CDI, on ne peut y voir que des avantages au moins pas de dégradation de la situation, par contre la tentation va grandir prendre l'exemple de PSA, assure M. par exemple, on est passé de 12000 employées à 4000 employé sur une période de 7 à 8 ans aujourd'hui, PSA, on retrouve un peu d'oxygène à du dynamisme de la vitalité et par conséquent a besoin et a besoin de créer, créer des emplois. Antérieurement, comme il avait besoin quand même sur une période assez longue d'ouvriers parce que, en général, le cycle de fabrication d'une voiture, et surtout ceux de sa mise sur le marché et de son succès sur le marché, c'est sûr, de or de 4 à 5 ans, donc il ne pouvait pas se permettent de faire des CDD, il faisait des CDI et au moment où les problèmes se posent avec la voiture se des plus qu'il fallait licencier les débats, les licenciements économiques étaient assortis d'avantages financiers assez considérable et d'un accompagnement important reclassements par l'je je prends le pari que la facilité et la commodité pour PSA, demain ce sera de faire du CD Chantier plutôt que du CDI, avec tous les inconvénients qui vont accompagner ces CD chantiers : pas de prime de préparer, de précarité, pas de licenciements économiques et pas d'accompagnement. La parole est à monsieur abouti, je vous en prie, le vrai risque, monsieur Touraine aujourd'hui, c'est que si PSA doit augmenter ses effectifs en Franche-Comté ou en Bretagne, si effectivement il doit faire des CDI pour une période courte, c'est qu'effectivement,

effectivement je, je, mais l'avis du gouvernement et de la Commission, sachant que dans le mot projet de croissance, une opération, ça peut être une mission, ça peut être un projet, ça peut effectivement être être marcher et je crois que la différenciation, il s'agit. Pas d'une généralisation de ces contrats parce qu'il y a des choses qui s'y adapter, d'autres pas, bande de la quincaillerie et construire un paquebot, c'est pas la même chose et il est bien évident que pour construire un paquebot pour construire un nouveau modèle, il y a des à-coups qu'on peut prévoir sur une certaine durée, et puis s'il y a récurrence de cette croissance, hé bien, il peut y avoir ensuite des CDI, je dirais des définitif, mais il y a, il y a des missions, les lignes, les marchés sont de plus en plus fluctuante des visibilités sont de plus en plus courte, aller dans des entreprises ont des PME de fabrication ou de services, même dans des entreprises de taille moyenne, demandez leur les délais de plantes charge qu'ils avaient il y a 20 ans, à niveau de niveau de production équivalent, les délais pour une charge qu'ils avaient il y a 20 ans et les délais qu'ils ont aujourd'hui les délais de visibilité des entreprises ont été divisés par 2, par 3 ou par 4 suivant les professions, vous avez de l'entreprise de plus de, de, de plusieurs centaines de salariés qui ont une vision de plan de charge qui ne dépasse pas la semaine, comment voulez-vous être flexible et vous adapter si vous n'avez pas des souplesses en matière de marché du travail, c'est pour ça que je, je dis il faut voir comment fonctionne vraiment nos activités, alors on peut être contre le fonctionnement des activités si l'mais à ce moment-là, si on n'a pas de réactivité d'entreprise elle disparaît et les employes et disparaissent donc je dire qu'on a besoin de la protection a besoin de garanties, mais on a aussi besoin je dirais d'une flexibilité qui permette de répondre aux conditions du marché et je n'ai pas l'ambition et nous ne pouvons pas transformer les conditions du marché, elles sont ce qu'elles sont.

affaiblir même le contrat à durée déterminée, parce que, avec le contrat à durée déterminée qui est assez difficile à rompre, il y a la prime de précarité ça été évoqué ici et là, ce serait le comble par ailleurs je voulais aussi verser au débat que on a déjà pas mal, 2 types de contrats différents le CDD d'usage : si on en fait le bilan, l'IGAS dit

on me dit que le cet amendement de repli que je défends ne serait quasiment pas recevable, mais en tous les cas, il a été reçu et qu'on me demande de le retirer parce que n'est pas évoqué dans ce projet de d'expérimentation, je regrette parce que, à la rigueur, on pourrait se dire, puisque vous n'avait fait aucune étude d'impact réel sur le nombre d'embauches possibles en vous prenant au mot voulait bien faire, nous, on a soulevé ici les graves dangers mais si on vous prend au mort, on peut se dire Banco à expérimenter et voyons Madame Bricq a évoqué l'expérimentation sur. 5 ans, donc ça existe dans notre loi, ça serait bien, des fois, de commencer à amorcer des hypothèses et d'en tirer les bilans d'ailleurs comme Hollande, il tire le bilan : ils vont revenir en arrière, parce que ça complètement foiré et je vais employer un terme, ça a été ça a été de la précarisation à l'intérieur des entreprises et aucune embauche de ce qui n'était pas dans l'entreprise on fait cette évaluation, moi je vous propose, dans un secteur qui, d'ailleurs Madame Bricq a évoqué, évoqué, le numérique et les Start-Up la tentons ça, faisons le bilan parce que nous savons que les contrats de projets peuvent avoir merci mon cher aujourd'hui, en tous les cas c'est évoquée. Merci mon cher collègue, la parole est à madame Cohen.

le recours aux contrats à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération mais on l'a dit, c'est complètement un glissement de langage, on parle de contrat à durée indéterminée donc indéterminé, ça a un sens, mais chers collègues mais on dit pour la durée de chantier ou d'une opération.

donc on va amplifier la précarité et on veut généraliser les choses, j'entends on me j'ai entendu dans cet hémicycle va positif pour l'entreprise pour la productivité et il y a eu l'exemple de prix de, de, de cadres de haut niveau mais ça veut dire que, en fait, les entreprises, je pense aux grands groupes, ils vont piocher et vont le prendre comme ça les arrange, comme ça les arrange un certain nombre, finalement de 2 salariés de haut niveau, mais il y aura pas que les salariés de haut niveau mais, chers collègues, c'est-à-dire qu'en fait on on est en train de construire un modèle de société où on prend les salariés comme des Kleenex, c'est-à-dire qu'on les utilise sur un contrat de travail qui est à une durée déterminée, et puis après, on a plus besoin, on les jette, mais enfin dans un pays où le taux chômage était énorme, où on voit que retrouver un travail après une période de chômage est extrêmement difficile, moi je n'entendent pas dans cet hémicycle, depuis que nous avons commencé à discuter une démonstration nous prouvons que ça va réduire le le le problème du chômage et que ça va aider il y a les élus salariés dans les entreprises, d'autant que toutes les autres barrières disparaissent petit à petit on fusionne les, les, les, les IRP on retire toutes les protections des des salariés, donc on est dans un tout, là on est dans une explosion de la précarité sous un couvert soi-disant de faire attention à l'entreprise, etc, et là ce que je trouve c'est que cet abus de langage est vraiment grave en ce sens où on du Nord nous nos concitoyens, on essaye de nous du temps du pain aussi au Parlement. Merci, ma chère collègue,

pour. Et contre. Qui s'abstient, ils ne sont pas adoptées, je mets au voile amendement 215 rectifier bis avec 2 avis défavorables qui est pour.

Pour cet amendement sur le contrat de croissance effectivement si j'ai bien compris peut être satisfait à travers l'évolution des choses, donc c'est bien volontiers que je le retire. Si mon cher collègue, et sur la maman demande 105 rectifié, il y avait une demande de retrait.

quant aux 206 j'ai entendu qu'il y avait un manque de précision sur le secteur concerné, donc je pense qu'on y reviendra, mais je retire également. Si ma chère collègue je vais suspendre la séance, nous avons examiné 37 amendements, ce matin,